La séance est reprise. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée contre toutes les fraudes aux aides publiques. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 3, précédemment réservé à l'article 3. Je suis saisi d'un amendement 95. C'est monsieur Verzelen qui nous le présente. Prenez le temps qu'il vous faut, cher collègue. Merci M. le Président. Je vais pas refaire les propos de la discussion générale. Nous sommes ici dans des articles, des éléments qui ont été votés dans le cadre de la PPL à l'Assemblée et au Sénat. Et il s'agit ici de renforcer les sanctions en cas d'abus de faiblesse. Je vous remercie. Merci. Quelle est l'avis de la Commission, M. le rapporteur ? Mes chers collègues, chers collègues Pierre-Jean Verzelaine, cet amendement reprend les amendements n°3 de madame Vogel et n°9 de la rapporteur de votre texte ici au Sénat au mois de novembre, madame Richard. Tous deux ont été adoptés par le Sénat lors d'examen de la proposition de loi, la vôtre, avec la vie favorable de la Commission et la vie de sagesse du gouvernement. Il vise, comme vous l'avez expliqué, à inclure dans la liste des pratiques commerciales interdites, le fait de subordonner la vente d'un bien d'un service à l'acceptation du démarchage téléphonique et à renforcer les sanctions encourues en cas d'abus de faiblesse liés au démarchage téléphonique. Ça sera naturellement comme un certain nombre d'avendements que vous présenterez, chers collègues, qui reprennent ni plus ni moins que votre proposition de loi qui a été votée ici à l'unanimité. Ça sera un avis favorable. Merci. Quel du gouvernement, Madame la Ministre ? Merci Monsieur le Président. Salut d'abord Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Donc cet amendement, Sénateur pardon excusez-moi, c'est d'avoir passé 12 ans dans une autre chambre. Je vous prie de bien vouloir excuser cette différence. Cet amendement que vous proposez Monsieur le Sénateur vise à interdire de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service au consentement du consommateur. à être démarché par voie téléphonique et à durcir les sanctions encourues lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance est commis à la suite d'un démarchage téléphonique. à cet amendement puisqu'il est en cohérence comme cela a été dit par monsieur le rapporteur avec la rédaction de votre proposition de loi sur le démarchage téléphonique. Je veux juste signaler que cette peine d'amende que vous portez ici à 20% du chiffre d'affaires est nettement différente de celle qui figure d'une manière générale dans le droit à la consommation qui est un niveau de 10%, donc qui sera important éventuellement de réaliser un travail d'affinage du degré de sanction, ce qui pourra être fait éventuellement en CMP. Avis favorable. Merci, je mets au voie cet amendement 95 avec deux avis favorables, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous passons ensuite à trois amendements identiques, le premier et le 41 défendu par monsieur Michaud. Oui monsieur le Président, le Président, Madame la Ministre, chers collègues, si l'article 3 prévoit déjà un ensemble de dispositifs, visant à renforcer la protection du consommateur, nous estimons qu'il faut encore aller plus loin en matière de lutte contre les fraudes et les arnaques de toutes sortes qui sévissent dans le secteur du démarchage à domicile. L'article L221-10-1 du Code de la consommation prévoit l'interdiction du démarchage à domicile non consenti. Mais dans les faits, nous le savons tous et toutes ici, les consommateurs ne connaissent pas vraiment l'existence de leur possibilité de matérialiser leur refus de recevoir des sollicitations commerciales à domicile. Nous souhaitons donc en complément cet article du Code de la consommation que le consommateur peut exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen à sa disposition et notamment par voie d'affichage. Enfin, notre amendement prévoit la caducité des contrats qui seraient inscrits en dépit de l'opposition des consommateurs d'être démarchés à domicile. Nous pensons donc que ces dispositions seront à même de protéger les consommateurs et de mieux lutter contre tous les types de fraudes pouvant exister. Je vous remercie. Cela fait plusieurs années que nous essayons d'encadrer le démarchage téléphonique et malgré ça, mes chers collègues, les sollicitations intempestives sont constantes et nous en sommes témoins tous les jours. Aussi, comme le propose du FC Quechoisir, nous pensons que le consommateur doit être en mesure d'exprimer son refus de recevoir des sollicitations à domicile par tout moyen à sa disposition et notamment par voie d'affichage. Enfin, il est essentiel de prévoir la caducité des contrats qui seraient souscrits en dépit de l'opposition des consommateurs à être démarchés à domicile. Trop souvent, en effet, de guerrelaces, certaines personnes se retrouvent engagées dans un contrat pour, entre guillemets, se débarrasser du démarcheur.

Oui, très rapidement, parce qu'il s'agit exactement du même amendement qui a été très bien défendu. Je se rappelais que c'est une proposition de l'UFC que choisir. Merci. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur ces trois amendements identiques. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Trois amendements identiques. Chers collègues, on a le groupe socialiste on va dire, présenté par notre collègue Michaud. le groupe communiste et les écologistes avec notre collègue Gontard. L'article en question du Code de la consommation interdit déjà le démarchage à domicile lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambigüe ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite. Il ne me semble pas nécessaire de préciser au niveau de la loi que le consommateur peut utiliser une affiche à cette fin. Surtout, la présomption de culpabilité que vous introduisez est très forte. Cela me semble induire des risques juridiques. Chaque entreprise qui aura vendu un bien au cours d'un démarchage à domicile devra prouver qu'elle n'était pas en tort. Mais comment apporter cette preuve ? Et comment les services pourront-ils absorber cette charge de contrôle ? Il vaut mieux renforcer les pouvoirs d'enquête et de sanction de la DGCCRF, comme l'a fait la Commission, et bien sûr faire en sorte que les consommateurs soient mieux informés de leur possibilité d'afficher le refus d'être sollicité à domicile. Madame la Ministre pourra certainement nous éclairer sur ce qui est mis en œuvre par la DGCCRF pour limiter ces abus. Ce sera donc un avis défavorable sur les trois amendements. je fais pourtant des efforts mais c'est douze ans qui m'ont marquée probablement. Messieurs les sénateurs, ces amendements identiques ont pour objet de renforcer la protection des consommateurs contre le démarchage à domicile. Ce n'est pas l'objet de la présente proposition de loi. Par ailleurs, la directive européenne dite Omnibus a d'ores et déjà renforcé la protection des consommateurs en matière de démarchage à domicile. Et je vous cite d'ailleurs ce que dit cette directive Omnibus qui indique que toute visite non sollicité d'un professionnel au domicile d'un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet il y a déjà une disposition qui est prévue. de points concernant le démarchage à domicile. Il y a d'ailleurs des dispositifs que vous pouvez mettre sur votre téléphone portable pour communiquer avec la DGCSERF sur un certain nombre de situations qui se présentent. Et la DGCSERF, bien sûr, établit un certain nombre d'enquêtes et établit des sanctions derrière. Donc, pour les raisons évoquées, avis défavorables du gouvernement sur ces amendements. Merci Madame la Ministre. Je mets au voie ces quatre amendements identiques, 41, 72, 114, avec deux avis défavorables, qui est pour, s'il vous plaît. Merci. Qui est contre ? Ils ne sont pas adoptés. Je vous remercie. Monsieur Verzelaine, vous nous présentez le 96, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il s'agit ici d'interdire aux professionnels de recontacter par téléphone un consommateur ayant exprimé son opposition. Merci. Merci. Quelle est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur ? Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, chers collègues Verzelaine. Je le dirai à chaque fois mais cet amendement permet d'introduire dans la PPL l'intégralité de votre proposition de loi votée à l'unanimité au Sénat et donc ça sera un avis favorable. Merci, l'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Je veux en premier lieu saluer tous les travaux qui ont été conduits par le Sénateur Verzelaine au travers sa PPL sur ce sujet qui intéresse beaucoup les Français. Le gouvernement est favorable à votre amendement puisque finalement cela permet aux consommateurs d'avoir la main sur son consentement pour empêcher un professionnel de le contacter à nouveau. et de mettre fin à l'appel. Cela nous paraît être deux excellentes choses. Cela nous permet de respecter la liberté des uns et des autres et notamment du consommateur. Un avis favorable. Merci. Je mets au voie cet amendement 96 avec deux avis favorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons ensuite à neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier défendu par monsieur Richard. C'est le 24. Vous avez la parole, cher collègue. Voici un amendement particulièrement important à mon sens. L'article 3 consacre le consentement préalable du consommateur à être démarché par téléphone. C'est dans le cadre du régime Optin dont on a parlé tout à l'heure. Dans la mesure où ce nouveau régime vaut pour tous les domaines économiques, ma question est la suivante. Pourquoi maintenir une interdiction sectorielle et tout particulièrement celle qui existe en matière de rénovation énergétique ? Le maintien de l'interdiction existante de démarche-âge téléphonique dans ce secteur et l'introduction envisagée d'une introduction à un autre secteur, ainsi même que l'extension de ces interdictions à d'autres modes de prospection commerciale, me paraissent présenter des risques sérieux de non-conformité avec les directives européennes concernées, lesquelles, comme vous le savez, prohibe les interdictions absolues. Un tribunal administratif, celui de Rennes, a décidé que l'interdiction de la prospection commerciale par voie téléphonique en rénovation énergétique était incompatible avec les objectifs d'une des directives européennes dont je viens de parler. DGCCRF d'ailleurs a mis en place une tolérance administrative vous le savez bien Madame la Ministre permettant aux entreprises d'appeler des consommateurs en rénovation énergétique s'ils ont donné leur accord préalable et on parle bien ici d'accord préalable donné dès lors L'application du nouveau régime de l'optin au secteur de la rénovation énergétique ne serait pour moi que la légalisation de la tolérance administrative en vigueur depuis trois ans. Je viens d'en parler. En outre, ces interdictions pour certains secteurs et modes de commercialisation me paraissent induire une vraie inégalité de traitement, une distorsion de concurrence. Elles sont aussi, à mon sens, susceptibles de

Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement propose d'introduire l'interdiction du démarchage domicile dans le domaine de la rénovation énergétique en cohérence avec l'extension prévue par la présente loi de l'interdiction des sollicitations commerciales sur ce secteur d'activité aux mails, SMS et réseaux sociaux. Nous le savons, le secteur de la rénovation énergétique concentre un très haut niveau de litiges de consommation et d'escroqueries réalisées en particulier sur des personnes âgées ou vulnérables. C'est la raison pour laquelle la prospection commerciale par téléphone dans ce domaine a été purement et simplement interdite par la loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et a lutté contre les appels frauduleux de juillet 2020. Mais le démarchage à domicile est encore plus intrusif et beaucoup plus dangereux pour le consommateur. Pour les associations de défense des consommateurs comme l'UFC que choisir, son autorisation par la loi à manière de rénovation énergétique rend possible la création de sociétés dont l'objet est exclusivement d'opérer des escroqueries des escroqueries à grande échelle visant des personnes Le consommateur finit par donner son accord à un achat qu'il n'aurait jamais effectué dans des conditions normales. Dans certains cas, le démarcheur peut parfois faire signer un faux document de renoncement à l'usage du droit à rétractation. Au-delà du préjudice pour les victimes et l'impératif de protéger les consommateurs, l'interdiction du démarchage à domicile pour la rénovation énergétique permettrait ainsi de mieux lutter contre les fraudes et malfaçons propres à ce type de protection commerciale. Merci, monsieur Laylek. Vous avez un amendement identique, le 51. Merci, monsieur le Président, madame la Ministre, messieurs les après le démarchage par téléphone, mail, SMS, réseaux sociaux, la question du démarchage à domicile dans le domaine de la rémunération énergétique pose des questions. J'ajoute que sur chaque présul 10 dont il est question, c'est 20 000 euros en moyenne par dossier. ce sont des personnes extrêmement vulnérables et souvent âgées. Et la DGCCRF, en même temps que l'UFC Cochoisir, alerte sur les démarcheurs et qui prétendent aider les victimes de fraude aux travaux de rénovation énergétique en se faisant passer eux-mêmes pour des délégués d'associations de consommateurs et nous appelle à légiférer sur cette question. Donc, pensons que c'est un amendement de bon sens. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. M. le Président Gontard, vous avez l'amendement identique 115. Oui, merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, M. le Président. C'est effectivement un amendement de bon sens puisqu'il s'agit du même amendement qui vise à interdire le démarchage physique pour lutter contre les arnaques aux travaux aux travaux de rénovation des logements, mais aussi à l'adaptation au vieillissement ou handicap de ces logements. On sait que ces démarches abusives, justement à la fois physiques, vont directement pour imposer des procédés, sont source de fraudes importantes. Je rappelle quand même que cette disposition avait été intégrée par l'auteur et le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. et que ça avait été jugé en s'appuyant sur une directive européenne qui du coup ne permettait pas justement cette disposition. Je rappelle que les États membres peuvent agir sur le motif d'intérêt public et il me semble que nous sommes bien dans ce cadre d'intérêt public, donc cette disposition pourrait tout

Oui, c'est un amendement identique. Il concerne le démarchage par mail. Le droit en vigueur prévoit déjà la règle de l'opt-out pour l'envoi d'emails de prospection à des clients et la règle d'opt-in pour l'envoi d'emails à des prospects. Concernant le démarchage sur les réseaux sociaux, la loi de 2023 dite « influencer » a introduit des mesures pour mieux encadrer le démarchage commercial effectué via les influenceurs et améliorer l'information des usagers. Le groupe RDSE considère que ces règles doivent d'abord être évaluées au regard de leur efficacité avant d'être améliorées. Il estime dès lors que l'interdiction sèche, introduite par l'article 3, pose le risque de préempter cette démarche. Merci. Madame la Présidente, qui défend le 52, monsieur Houpert, monsieur Richard ? Il est défendu... Il est défendu, je vous remercie. Le 108 n'est pas défendu dans l'hémicycle. Nous passons 54 et c'est M. Cannevet Merci M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues. Il s'agit de permettre aux entreprises disposant d'un label de qualité de pouvoir néanmoins mener des actions de prospection commerciale. Merci. Quel est l'avis de la Commission, M. le rapporteur Merci Monsieur le Président. Alors on va procéder en trois ou quatre étapes concernant l'amendement numéro 24 de nos collègues André Reichardt. Par votre amendement, chers collègues, vous revenez sur l'interdiction du démarchage téléphonique dans la rénovation énergétique issue de la loi Nijlène et sur son extension au secteur de l'adaptation des logements. Ne rejoint pas tout le débat de 2020. Ces interdictions sectorielles sont justifiées car elles permettent de cibler des entreprises potentiellement frauduleuses qui jouent sur les aides distribuées par l'Agence nationale de l'Habitat. Je rappelle que selon la DGCCRF, cette interdiction du démarchage téléphonique pour les rénovations énergétiques n'est toujours pas respectée près de 5 ans après la loi Nechelen. Les amendes de la DGCCRF pour non-respect de cette interdiction s'élèvent tout de même à 4,4 millions d'euros en 2023. Je rappelle aussi que certaines entreprises malhonnêtes se rabattent sur la prospection par voie électronique pour compenser le fait que nos concitoyens décrochent de moins en moins leurs téléphones face à un numéro inconnu. En plus d'être inondés d'appels, nous recevons de plus en plus de messages personnels par mail, voire sur des messageries instantanées. N'allons pas au-delà du vote du Sénat le 14 novembre dernier et n'oublions pas que les secteurs de la rénovation énergétique et de l'adaptation de logements concentrent les fraudes. Ce sera donc une demande de retrait, chers collègues, ou un avis défavorable. Concernant les amendements identiques 40, 71, 115 de nos collègues Michaud, Guet et Gontard. Mes chers collègues, vous avez raison. Le démarchage à domicile abusif est un vrai fléau qui peut générer des abus de faiblesse. Mais il me semble qu'il y a un sujet de conformité aux droits de l'Union européenne. La directive dit Omnibus précise que si les États membres peuvent prendre des dispositions renforçant la protection du consommateur dans le cadre de visites non sollicitées ou non souhaitées, c'est l'objet de vos amendements, ces dispositions doivent être proportionnées. Cela ne serait peut-être pas le cas en cas d'interdiction totale. Néanmoins, Madame la Ministre, est-ce qu'une interdiction fondée sur l'intérêt public liée à la lutte contre la fraude permettrait d'être en conformité avec le droit de l'Union européenne ? Il est vrai qu'en matière de rénovation énergétique, le taux d'anomalie des établissements contrôlés par la DGCCRF s'établit à 51%. Il y a un vrai enjeu de fraude. C'est la raison pour laquelle je demande sur ces trois amendements la vie du gouvernement. Pour les amendements identiques numéro 37 47 52 et 52 puisque le 108 n'a pas été défendu je crois. Sur le fond je pense qu'au contraire l'interdiction de la prospection commerciale par voie électronique dans le domaine de l'adaptation des logements est pertinente car de nombreux professionnels malhonnêtes se reportent sur les emails et messages sur les réseaux sociaux pour contourner l'interdiction du démarchage téléphonique dans ces secteurs qui n'est toujours pas bien respecté comme je le rappelais précédemment. Je précise et je l'ai dit au cours de la discussion générale que la publicité est très différente de la prospection commerciale. Quand on parle de prospection commerciale par voie électronique, ne sont visés que les messages personnels sur les réseaux sociaux par mail ou sur un service de communication interpersonnel. On ne va bien évidemment pas interdire à une entreprise de communiquer sur les réseaux sociaux, ni de faire de la publicité. Il faut être très clair, ce sont deux choses très différentes. ne sont visées que les messages personnels que l'on peut recevoir via les réseaux sociaux, mais pas les publications en ligne sur ces réseaux sociaux. J'ai régulièrement des amis qui sont chefs d'entreprise dans le bâtiment, qui mettent des photos de leur réalisation et qui les mettent sur un poste FB. Ça ne sera pas interdit. La publicité non plus. On parle de messages personnels. Donc sur ces trois amendements, ça sera une demande de retrait ou à défaut, en avis, défavorable. Et enfin, pour l'amendement 54 de notre collègue Cannevet, je crois, Je crains qu'une telle exception ne complexifie le contrôle et n'entraîne des contournements de la part d'entreprises malhonnêtes. Vous connaissez mon obsession pour la simplification. Plus c'est simple, plus c'est facile à contrôler, plus c'est facile à sanctionner. Nous avons énormément de remontées de fraudolabels, notamment le RGE, dans le cadre de cette PPL. En outre, l'interdiction du débarchage par voie électronique poursuit un objectif simple, la protection des consommateurs. Ça sera donc un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Les avis du gouvernement, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président. Un grand nombre d'amendements déposés qui concernent tout le sujet de la rénovation énergétique en ce qui concerne le premier 24 de Monsieur Richard. Plusieurs points, un premier que vous avez d'ailleurs évoqué en indiquant que la DGCCRF a mis en place une tolérance administrative qui permet aux aux entreprises aujourd'hui d'appeler les consommateurs en rénovation énergétique s'ils ont donné leur accord préalable. Et effectivement, le consentement préalable du consommateur à être appelé ne peut être assimilé à de la prospection commerciale téléphonique dans la mesure où il y a cet accord. Deuxième point, c'est qu'en ce qui concerne les sollicitations par voie numérique, nous avons énormément de fraude à la rénovation énergétique et ça a été rappelé par un certain nombre de sénateurs qui se sont exprimés et à tout ce qui concerne l'adaptation au logement avec de nombreuses tentatives et nous avons tous des exemples sur les territoires d'abus de faiblesse envers des populations qui sont particulièrement vulnérables donc il nous faut protéger. Pour l'ensemble de ces éléments je donne un avis défavorable à cet amendement 40. Nous avons ensuite les amendements 37, 47 et 52, qui vise à la suppression de l'interdiction de démarchage par courrier électronique, SMS et réseaux sociaux en ligne pour certains secteurs déterminés, notamment la rénovation énergétique. pour les mêmes raisons que ce qui est évoqué en matière de fraude vis-à-vis d'un grand nombre de dispositifs de fraude dont nous dont nous avons été les uns et les autres alertés. Donc il est important de protéger les populations fragiles et préciser par ailleurs que la plupart des artisans et entreprises honnêtes du secteur n'ont pas forcément besoin de recourir à de telles méthodes de démarchage pour se constituer une clientèle. Les amendements 47 et 52 sont un peu de nature différente puisqu'ils visent à la suppression de l'interdiction de démarchage par courrier électronique, SMS et réseaux sociaux pour les secteurs déterminés dont nous avons parlé et là pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées fraude à la rénovation énergétique et adaptation du logement. avec un grand nombre de démarchages intempestifs, également avis défavorables et pour les mêmes raisons ce sera également un avis défavorable sur le 54. Madame ministre, si je comprends bien, sur les trois amendements identiques 40, 71 et 115, vous avez donné un avis défavorable. Très bien. Et sur les 37, 47 et 52, aussi un avis défavorable. Est-ce que vous suivez l'avis de la ministre sur le 40, 71 et 115 ? Très bien. Merci. Je vais donc mettre au voie

à quel point il y a un sujet sur les démarchages à domicile, parce que c'est le vecteur majeur d'amorce des fraudes. Je le dis parce que je n'ai pas bien compris les motivations, madame la ministre, donc si vous pouvez, j'allais dire, nous approfondir. Parce que dans la directive européenne, moi je cite, Lorsque ces restrictions au démarchage commercial donc sont adoptées pour des motifs autres que la protection des consommateurs tels que des motifs d'intérêt public ou des motifs liés au respect de la vie privée des consommateurs protégés par l'article 7 de la charte, elles ne relèvent pas du champ d'application de la directive, elles ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Ça, c'est la directive Omnibus et c'est le contenu même du texte. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. il faut traiter la problématique du démarchage à domicile. On évoque un certain nombre de textes. Quand je regarde les textes, ce n'est pas ce qu'il est indiqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Pour explication de vote. merci Monsieur le Président. Moi je voudrais naturellement revenir sur l'amendement 24 et dire au rapporteur qu'autant je le remercie pour son ouverture d'esprit et le travail qu'il a fait, autant je voudrais juste lui rappeler qu'on n'est plus dans la même situation que lors de la PPL Negelen que j'avais l'honneur de rapporter à l'époque. Maintenant on est en opt-in, c'est-à-dire on décide d'accepter ou non le démarchage et donc dans ce cas-là qu'on me dise pourquoi il y a lieu d'interdire en plus. Il suffit que la personne se... décide à ne pas accepter un démarchage pour que la situation soit réglée. Pourquoi une interdiction ? ? Ensuite, pour madame la ministre, vous nous dites qu'il y a trop de fraude dans le domaine de la rénovation énergétique. Je voudrais juste vous rappeler que cette interdiction existe déjà depuis un moment. Et s'il y a des fraudes, c'est que manifestement on passe outre l'interdiction. A telle enceinte d'ailleurs que le tribunal administratif, puis une cour d'appel, ont dit qu'il faut en tenir compte de cet accord. Et donc on voit bien là qu'il y a une mutation qui se fait parce qu'effectivement on n'arrive pas à juguler la fraude. vous nous dites qu'il faut sanctionner ceux qui effectivement ne respectent pas, mais il y a le RGPD pour ça, il y a le RGPD pour ça qui sanctionne très directement ceux qui effectivement ne tiennent pas compte de la volonté des uns et des autres. Donc je suis obligé de vous dire que moi je maintiens vraiment cet amendement et je ne comprends pas comment à partir du moment où le démarchage n'est possible, téléphonique, Et naturellement, son ouverture numérique me paraît complique, excusez-moi mes chers collègues, me paraît complètement fou, cette interdiction à partir du moment où obligatoirement pour être démarché, il faut donner son accord. Pourquoi faut-il en plus dire dans tel secteur, tel secteur, tel secteur, ce sera interdit complètement ? Franchement, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui me passe au-dessus de la tête,

les explications de Madame la Ministre. Un, tout le monde dit, sur la rénovation énergétique, les entreprises vertueuses, et il y en a, il faut le redire, elles n'ont pas besoin de faire du démarchage à domicile. Tout le monde se met d'accord. Bon. Deuxième question. Les fraudeurs, eux, ils ont besoin. Et en réalité, je l'affirme ici, tous ceux qui font du démarchage s'adressent à des personnes âgées ou vulnérables. Et d'ailleurs, la question du consentement ou pas, ils en ont cure parce qu'ils vous feront signer un papier en même temps qu'un devis. Je rappelle, 20 000 euros en moyenne, le préjudice, c'est quand même extrêmement conséquent. Et tout le monde dit, tous ceux qui réalisent du démarchage à domicile sur cette question-là, potentiellement en tout cas sont des fraudeurs. Et la troisième chose, c'est qu'on sait que, à juste raison, le droit européen nous le permet si c'est d'intérêt public. Et pour le coup, interdire que des personnes vulnérables se fassent avoir par des escrocs, nous pensons, je pense à peu près, tous sur ces bancs, que c'est d'intérêt public. Donc à un moment donné, On ne touchera pas les entreprises vertueuses. On va permettre aux escrocs de ne plus pouvoir réaliser la chose et en vérité protéger les consommateurs et les consommatrices. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette question-là. Et pardon, mais le démarchage, en plus ailleurs, on pourra en débattre. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose... Je l'ai subi. Bon, il est tombé sur la mauvaise personne, quelqu'un qui s'est fait passer pour un AGVDF, et qui, en réalité, était quelqu'un en train de vouloir me vendre un contrat d'un énergéticien alternatif. Alors bon... Il a été reçu. Mais sérieusement, aujourd'hui le démarchage, c'est ça ! Mais sérieusement, c'est ça ! Donc on devrait pouvoir se mettre d'accord, c'est un intérêt public et l'intervient. Je vous remercie, M. le Président. Merci, je suis obligé de vous couper le courant, M. Gué, désolé. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Pour répondre à quelques-unes des interventions, je pense que sur les différents bancs, chacun constate qu'il y a un certain nombre de fraudes. Je crois qu'il y a un accord sur ce sujet. Alors finalement, est-ce que quand on constate qu'il y a des fraudes et qu'on regrette qu'il n'y en ait de trop, on ne peut que le regretter, est-ce qu'il faut au contraire élargir le dispositif, ouvrir le dispositif ? Parce qu'effectivement, si nous l'ouvrons, probablement qu'il y aura encore plus de fraudes. Voilà, donc à cette question-là, moi je ne souhaite pas ouvrir plus parce qu'effectivement, cela conduirait probablement à avoir plus de fraudes. Par ailleurs, je rappelle, M. Richard, et vous l'avez vous-même dit, qu'il existe une tolérance administrative aujourd'hui que la DGCC-ARF a mis en place et qui permet finalement d'avoir un contact, le cas échéant, sur ces sujets de la rénovation énergétique. également dire que Moi je connais un certain nombre de personnes qui font faire des travaux de rénovation énergétique et qui n'ont pas besoin forcément d'être sollicités par du démarchage. partout sur les territoires des entreprises qui sont verteuses, et vous l'avez vous-même dit, qui sont honnêtes, qui sont connues du territoire, qui sont des acteurs locaux et qui n'ont pas besoin de disposer d'un certain nombre de dispositifs de démarchage. Voilà. C'est en tout cas pour ces raisons que j'ai mis des avis défavorables sur ces amendements. Merci. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je vais répondre à notre collègue le Sénateur Reichard qui m'a demandé plus de précisions sur mon explication, mes commentaires sur son amendement. Là, je voudrais parler du message politique envoyé. Effectivement, on a la loi de notre collègue Pierre-Jean Verzelaine qui, quelque part, règle le problème d'une manière assez forte et assez large. Mais il ne vous a pas échappé dans le commentaire que j'ai fait que cette loi, moi j'ai dit neiglène, c'est peut-être néglène, mais bon, c'est neiglène, que cette loi neiglène n'est pas respectée encore. 4,4 millions d'euros d'amende, rien que pour l'année 2023, pour non-respect de cette loi. Quelle serait la réaction des entreprises fraudeuses si le message qu'on envoyait c'était de dire, il n'est plus dorénavant interdit de faire ce genre de choses par rapport à la loi Négelène, puisqu'on l'a fait, entre guillemets, passez-moi l'expression, sauter au Sénat. Bah c'est qu'aujourd'hui c'est permis, puisque c'est plus interdit. puisque ce n'est plus interdit. Donc très mauvais message politique et moi je vous parie. que c'est plus 4,4 millions d'euros derrière. C'est beaucoup plus et beaucoup plus de fraude et beaucoup plus de tentatives de fraude. Donc on ne peut pas envoyer ce message politique là de dire on a supprimé l'interdiction pour ce genre d'entreprise de faire ce genre de démarchage. Donc voilà, moi je pense qu'il y a ce qu'on vote et il y a la portée de ce qu'on vote et qu'il est très important qu'on en tienne compte, chers collègues. Donc je maintiens mon avis défavorable. la vie de madame la ministre. En réalité je suis d'accord avec vous dans ce que vous dites, c'est à dire que vous dites que des entreprises, et c'est une majorité des entreprises, qui font un très bon travail n'ont pas besoin de démarchage et d'ailleurs elles n'en font pas, c'est même souvent elles qui sont démarchées donc elles n'en ont pas besoin. On sait par contre que ce sont des entreprises qui elles posent problème, qui vont faire du démarchage et en réalité on sait très bien que quand il y a démarchage derrière Il n'y a pas qu'à 100% de fraude, mais on va dire qu'il y a une très grosse proportion de fraude. Donc évidemment qu'on a besoin d'encadrer. Et donc vous faites le même constat en disant, du coup, on ne fait rien. Et du coup, j'avoue ne pas comprendre. Madame la Ministre, après je clôturerai la discussion. Oui, juste vous dire que ce que vous évoquez est déjà prévu par la directive Omnibus, et j'ai eu l'occasion de le dire, qui a déjà renforcé la protection des consommateurs en matière de démarchage Donc si vous voulez, ce que vous appelez finalement est satisfait. Merci, je mets au voie cet amendement 24 avec deux avis défavorables qui est pour qui est contre, il n'est pas adopté. Je mets au voie trois amendements identiques 40, 71, 115, avec deux avis défavorables, qui est pour ? Ce qui est contre, Ils ne sont pas adoptés. Ensuite, trois amendements identiques, 37 47 52 avec deux avis défavorables qui est pour ? Personne, d'accord. Qui est contre ? Pardon, je ne vous ai pas vu. Pardon. Qui est contre ? Ils ne sont pas adoptés et l'amendement 54 est retiré, M. Cannevet. Nous passons ensuite au 88, M. Verzelaine, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes au cœur de l'intérêt du texte, en tout cas en ce qui concerne le démarchage téléphonique qui va être voté ce soir, c'est-à-dire le basculement de l'optaout à l'optin. L'optaout, nous sommes pour l'instant toujours dans ce cadre-là, ce qui veut dire que chaque Français, nous sommes tous considérés comme étant consentants pour être démarché téléphoniquement. C'est d'ailleurs ce qui explique depuis un moment que toutes les adaptations ont fonctionné, nous pourrons constater, plus que moyennement. Donc le basculement à l'optin, c'est le fait qu'une entreprise ne puisse nous appeler qu'à la condition que nous ayons obtenu son consentement. Et nous précisons dans cet amendement, enfin je précise, que le consentement de nos têtes libres, spécifique, éclairé, univoque et révocable. Simplement, ça veut dire quoi ? C'est plus une page pré-remplie et on coche en bas « ok », c'est à nous de compléter la page, c'est à nous de mettre nos coordonnées téléphoniques. Et le cas où nous serions appelés, dès que nous disions « stop », l'entreprise est obligée d'arrêter. Voilà la précision qui est apportée dans cet amendement. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous pouvez présenter les 89 dans la foulée ? Je crois qu'ils sont très proches. Oui, Monsieur le Président, il s'agit ici de préciser qu'il incombe à l'entreprise de prouver qu'elle a bien recueilli le consentement du consommateur pour être démarché. Merci. M. le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Favorable sur les deux amendements, M. le Président. Merci, Mme la Ministre. À l'avis du gouvernement. merci, M. le Président. Là, on est au cœur, finalement, du dispositif de cette PPL avec la définition du consentement et donc avis favorables sur ces deux amendements puisque vous le définissez de manière beaucoup plus précise et cela nous paraît très important. Merci Madame la Ministre. Je mets au voie l'amendement 88 avec deux avis favorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Il a adopté. Je mets au voie l'amendement 89 avec deux avis favorables. C'est le même vote ? C'est le même vote. Nous passons ensuite au 23, Monsieur Rechart. Vous avez la parole pour le défendre. Le 23, rectifié. Bisse. Le principe de l'exception n'est pas remis en cause par la PPL que nous examinons. Le débat concerne uniquement le périmètre ou les modalités de cette exception. Je pense, ainsi que les cosignataires de l'amendement, qu'il faut absolument libéraliser l'exception client et permettre aux professionnels d'appeler leurs clients pour leur proposer tout produit ou service qu'ils commercialisent. La protection du consommateur est assurée par l'ERGPD, lequel garantit un droit d'opposition à la conservation et l'utilisation des données à caractère personnel. Il ne faut naturellement pas la rendre encore plus stricte, cette exception client, bien au contraire. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission de ce rapporteur ? Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, chers collègues, André Reichardt. Je mettrai un avis favorable sur votre amendement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il me semble justifié de libéraliser cette exception client. Ne pas la restreindre au seul contrat en cours liant directement le professionnel au consommateur, comme l'ont fait les députés dans le cadre de l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi de notre collègue Verzelen. On ne met pas en cause par votre amendement Le régime d'optin de Monsieur Verzelen ? Pas du tout. Par contre, on permet aux entreprises, par rapport à leurs fichiers clients, à qui on va déjà imposer le système d'optin. On leur permet d'étendre les propositions qu'ils peuvent faire à leurs clients. À leurs clients. Et donc on respecte l'exception client dans ce fait-là. Donc un avis favorable à cet amendement. Merci Madame la Ministre, qui est l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Donc votre amendement prévoit que le professionnel peut démarcher par téléphone un client pour lui proposer tout produit ou service qu'il commercialise. Donc c'est une extension. Alors tout d'abord, ce qui me paraît un petit peu difficile, c'est la notion de client qui paraît trop vaste et non définie juridiquement. C'est un point. puisque cela veut dire ici qu'un professionnel pourrait démarcher de façon illimitée un consommateur dont le contrat a pourtant pris fin. Le deuxième point, et c'est là peut-être une question de rupture d'égalité, Puisqu'un tel amendement accorderait un avantage supplémentaire à une entreprise d'une certaine taille qui peut disposer d'un éventail de produits par rapport à une entreprise de plus petite taille qui n'a pas forcément une diversité de produits de cette nature. Voilà, donc j'y soulève quelques difficultés. Pour autant, j'entends ce que vous avez dit et je vais sortir de ma fiche. Je vais émettre un avis de sagesse.

Si je prends des groupes comme des grands énergéticiens avec des dizaines, des fois des centaines de filiales, est-ce que l'entreprise, c'est bien l'enseigne avec laquelle j'ai contracté qui est un sirène, ou est-ce que c'est avec l'ensemble de la panoplie du groupe ? Voilà, j'aimerais aussi que les choses soient précises et qu'on se limite bien à l'entreprise et l'enseigne et le sirène en tant que tel. Merci. Merci. Cher collègue, je mets au voie cet amendement. monsieur Houpert, vous vouliez la parole ? Je vous la donne. Monsieur le Président, Madame la Ministre, monsieur le rapporteur, vous aimez la simplification. Je pense que cet cet amendement simplifie les choses. Et si on se met à la place des entreprises, une entreprise qui a des contrats avec un client n'a pas intérêt à harceler le client à tout moment. Merci, je mets au voie cet amendement 23 avec un avis favorable. de la commission à l'avis de sa geste du gouvernement qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous passons ensuite à un amendement et un sous-amendement. L'amendement est le 91 défendu par monsieur Oui monsieur le Président, cet amendement précise que le consommateur peut être appelé en dehors des jours horaires et fréquences prévues par le décret si ce dernier a donné son consentement au professionnel faire l'entreprise pour être contracté à une date et à un horaire spécifiques. Monsieur Richard, vous avez sous-amendé cet amendement, c'est le 146. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je l'ai effectivement sous-amendé simplement par, je dirais pragmatisme, souhait de simplifier cet amendement qui me paraît aller dans le bon sens. Vous le voyez, plutôt que de préciser comme le dit l'amendement 91, si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés et qu'il peut l'établir, je propose de remplacer simplement si le consommateur il consent explicitement. C'est beaucoup plus simple, ce n'est pas une usine à gaz. Imaginez-vous s'il fallait effectivement que le consommateur consente en indiquant précisément quel jour il souhaite être appelé, il faut l'appeler pour savoir quel jour, enfin, Je pense qu'il faut être très simple dans ce dossier. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Votre avis sur l'amendement et le Merci, monsieur Merci, monsieur le Président, madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, sur l'amendement de notre collègue Pierre-Jean Verzelaine. On est dans la lignée des amendements de notre collègue, auteur de la PPL Interdiction. Donc, je mettrai un avis favorable. Sur le sous-amendement 146 de notre collègue André Raichard. Vous savez quel est mon acharnement sur la simplification, quel que soit le dispositif, et votre amendement vise à simplifier le dispositif tout en protégeant, et nous y avons prêté attention, tout en protégeant le consentement du consommateur. Ça sera également un avis favorable. Merci Monsieur le Président. Il s'agit ici de permettre Merci Monsieur le Président. Il s'agit ici de permettre aux consommateurs d'être appelés en dehors de cadre prédéfini à une date et à un horaire précis pour répondre à un besoin ponctuel voire urgent et tout ce qui participe à la liberté. et à donner de la latitude et à répondre aux enjeux des consommateurs va dans le bon sens. En ce qui compte, ça c'est pour l'amendement 91 donc un avis favorable. Quant au sous-amendement, il retire ici en fait le fait de préciser la date et l'horaire sur lequel le consommateur souhaite être pour autant ça me paraît important qu'il puisse choisir la plage horaire qui lui convient et c'est ce que vous retirez ici si je comprends bien en travers votre amendement donc je mettrais plutôt un avis défavorable parce qu'il me paraît important que le consommateur puisse participer à choisir sa date et son horaire. Donc avis défavorable sur le sous-amendement. Merci Madame la Ministre. Je mets au voie le sous-amendement 146 avec un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour Qui est contre ? Le sous-amendement est adopté. Je mets ensuite au voie l'amendement 91 avec un avis favorable de la Commission. Est-ce que vous maintenez votre avis favorable Madame ? la ministre défavorable. Donc, je répète, un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre l'amendement sous-amendé et adopté. Nous passons ensuite au 92. Monsieur Verzelen, vous avez la parole. Monsieur le Président, il est précisé ici que lorsqu'il recueille les données téléphoniques, le professionnel doit informer le consommateur, en l'absence d'un contrat en cours, que toute sollicitation suppose qu'il ait donné son consentement. Je remercie. Favorable, M. le Président. – Madame la Ministre, favorable aussi. Je mets au voie cet amendement 92 avec deux aides favorables, qui est pour, qui est contre et l'a adopté. Nous passons ensuite à cet amendement et quatre sous-amendements. Le premier et le 22, il est défendu par M. Pla, vous avez la parole. territoires. Le dispositif d'optin proposé par l'article 3 risque de faire disparaître une activité essentielle pour les territoires ruraux, consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, sur l'ensemble du territoire. Déjà que les populations qui habitent en zone rurale éprouvent un puissant sentiment d'abandon lié à la fracture numérique médicale et à l'éloignement des services publics, elle en sera amplifiée par cette disposition. Bien sûr, j'entends et je partage l'exaspération de nombreux Français face au démarchage téléphonique abusif. Mais cela ne concerne pas la livraison alimentaire à domicile qui convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d'épicerie particulièrement larges aux habitants des zones rurales éloignées des centres commerciaux et sans possibilité de mobilité. Alors qu'une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérantes dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle, dans la mesure où les clients de ces entreprises disposent rarement des ressources qui permettent de donner leur consentement. Un autre modèle est impossible à mettre en place dans des délais si courts. C'est pourquoi il convient d'examter le secteur alimentaire de l'interdiction absolue. Cette spécificité alimentaire a été reconnue lors de l'examen de la proposition de loi dédiée au démarchage téléphonique à l'Assemblée nationale. Et en fait, je terminerai parce que cette interdiction est mal perçue par les acteurs qui sont très peu nombreux de la distribution agroalimentaire. Ils sont quatre. Parce qu'en voulant sanctionner une grande majorité d'entreprises qui abusent du démarchage téléphonique et malhonnête ont puni une minorité qui respecte les principes mêmes de la loi sur le démarchage téléphonique. Merci. En déposant cet amendement, j'ai tenu compte évidemment de notre vote unanime intervenu ici contre le démarchage téléphonique abusif. J'ai tenu compte aussi des conditions apportées à l'Assemblée nationale pour exclure cette interdiction les activités liées à l'alimentaire. Et en déposant cet amendement, j'ai considéré aussi la situation particulière de nos populations vieillissantes isolées dans nos campagnes. Je l'ai fait en sachant que ces personnes en ont aussi assez d'être harcelées par téléphone, mais dans le même temps, ces personnes ont besoin d'être livrées notamment en produits congelés. Je l'ai fait aussi en conscience et en sachant que ces entreprises qui les desservent ne sont pas forcément des entreprises frauduleuses. Alors bien entendu, il ne s'agit pas avec cet amendement de multiplier les exceptions. Je connais l'opposition qui pourrait nous en être faite. Mais depuis le débat qui s'est prolongé ce matin en réunion de commission, il me semble qu'il est raisonnable. de prendre acte des propositions de sous-amendements qui ont pu intervenir depuis et qui visent à limiter la dérogation d'interdiction totale de démarchage téléphonique aux seuls denrées alimentaires surgelées et tout ça pour une durée limitée, ce qui veut dire qu'en limitant les choses dans la durée et en pouvant les circonscrire aux seuls denrées alimentaires surgelées, nous ne somberons pas dans une dérive inflationniste – passez-moi l'expression et c'est une manière de tenir compte de la réalité vécue également dans nos territoires. Merci de votre attention. l'exposé que vient de faire notre collègue Gérard Lahellec, car il faut penser aux territoires ruraux, il faut penser aussi à ces opérateurs économiques qui sont qui promeuvent les produits de nos territoires et qui permettent justement à une clientèle, je dirais, éloignée des distributeurs, des centres commerciaux, de pouvoir être provisionnés en produits de première nécessité. Et je me rappelle que la délégation sénatariale aux entreprises s'est rendue chez Tirier et combien nous avions pu admirer l'excellence de travail de cette entreprise. Et je dirais, quand on est dans la lutte contre la fraude, quand on examine un texte relatif à la lutte contre la fraude, on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même registre que l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur ce secteur-là. exposé Gérard Lélech, Moi, je dis aussi qu'il faut que, si l'on veut absolument empêcher ces acteurs de travailler, il faut leur donner du temps. Si l'on leur donne du temps, je pense qu'on va mettre en péril un certain modèle économique d'entreprise. Et nous, en Bretagne, qui sommes une région particulièrement portée sur l'agroalimentaire, nous savons bien combien il est important que les coopératives puissent effectivement desservir leurs adhérents. On voit bien que si un coup d'arrêt est mis à la capacité de ces entreprises de pouvoir desservir les clients, nous allons en devant de difficultés. Vous remercie. Monsieur Chassin, vous nous présentez l'amendement identique 101, s'il vous plaît. plaît. Oui, je vais quand même le présenter. Effectivement, mes collègues viennent de s'exprimer et c'est le même amendement. Cet amendement a pour objet d'exhanter le secteur alimentaire de l'interdiction totale de démarchage téléphonique. L'exaspération partagée par de nombreux Français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu'il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés d'épicerie, particulièrement, ça a été dit, aux habitants des zones rurales. Et ça a été dit aussi, une large partie de cette population souffre de fractures numériques, donc cette spécificité alimentaire a été reconnue lors de l'examen de la loi de proposition dédiée au démarchage téléphonique à l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Monsieur Grosvalet, vous nous présentez le 111. Il est défendu. Monsieur Buie, le 129, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors ces sept amendements identiques sont sous-amendés par quatre sous-amendements identiques. Le premier n'est pas défendu. Le second, c'est le 160, c'est M. Bourgois. M. Chaz, allez-y, excusez-moi, je ne vous avais pas vu, M. le Président. vu, M. le Président. Merci, M. le Président. Ce sous-amendement, effectivement, a pour effet, comme l'a précisé Gérard Laleck, de réduire encore la portée de l'amendement, de réduire aux produits surgelés uniquement et de réduire dans le temps à 60 mois son effet, ce qui pourra permettre aux entreprises de pouvoir se préparer à une nouvelle condition, sans difficulté ou en tout cas avec plus de facilité. Je crois que je veux dire ici que nous sommes tous sensibles à la problématique du démarchage. Par cette dérogation limitée dans le temps, on permet finalement à un secteur d'activité de pouvoir s'adapter dans les meilleures conditions sans remettre en cause la finalité de la loi de la loi qui on a tous voté. Merci, M. le Président. Ce sous-amendement vise à limiter la dérogation d'interdiction totale de démarchage téléphonique au seul rang alimentaire surgelé, et tout ça pour une durée limitée à 60 mois. Voilà la proposition. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, mes chers collègues. Je vais procéder en deux parties différentes et distinctes. J'y suis obligé, puisque les amendements, je procéderai à l'avis de la Commission.

concernant les amendements qui ont été débattus en commission. Je pense que vous l'avez tous compris, je ne suis pas favorable à la multiplication des exceptions à l'encadrement du démarchage téléphonique introduit par notre collègue Pierre-Jean Verzelaine. Et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que la moindre réception provoque une brèche. Une brèche provoque une volonté de contournement et donc une volonté de fraude. Soyons fidèles au vote à l'unanimité du 14 novembre dernier de la proposition de loi de notre collègue Pierre-Jean Verzelaine. Nous étions alors tous d'accord pour encadrer le démarchage qui exaspère les Français, vous l'avez tous dit, sans créer d'exception. Aucune. Sur le fond, l'interdiction du démarchage téléphonique sans consentement du consommateur n'empêchera pas les entreprises de travailler. Je rappelle qu'il existe une exception client, dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous venons d'ailleurs de libéraliser grâce à l'amendement de notre collègue André Reichard. L'optime ne signifie pas la fin du démarchage téléphonique, mais simplement du démarchage non sollicité. Les exceptions vont complexifier les contrôles. surtout générer des comportements fraudulés, une entreprise pourra se justifier à posteriori comme elle le souhaite, surtout si son activité est diversifiée. Donc vous comprendrez que c'est un avis défavorable sur l'ensemble des amendements et c'est un avis de la Commission. mon avis sur les sous-amendements. Trois points. Le premier. C'est une question de respect. Respect du travail de notre collègue Respect du travail de la rapporteure Olivia Richard qui ont travaillé, qui ont fait des auditions, qui sont allées à la rencontre des usagers, des entreprises et qui nous ont proposé une proposition de loi qui correspond à l'attente des Françaises et des Français. interdire définitivement, totalement le démarchage illicite qu'on subit tous, hein, moi j'en ai encore eu un tout à l'heure avant de revenir ici, respectant le travail qui a été fait. Le respect de la parole donnée. Nous nous sommes engagés, nous avons donné notre parole le 14 novembre dernier, devant tous les Français, ça a été salué par tous les médias le lendemain, que nous supprimions cette plaie des appels intempestifs. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne partage pas du tout vos paroles, mes chers collègues. On n'interdit pas les entreprises de travailler l'exception client qu'on a encore élargie avec l'amendement du collègue Reichardt. dire aujourd'hui que les clients qui sont dans les territoires ruraux ne pourront plus bénéficier des services, parce qu'on peut appeler ça un service, des services qui leur sont apportés, c'est faux. L'exception client donne toute largeur, toute possibilité, étendue par l'amendement du collègue Reichard, de continuer d'être appelé, livré, de la même manière qu'ils le sont aujourd'hui. Les clients qui ne le sont pas et qui souhaitent être livrés ont toute la possibilité, moi je veux bien qu'on parle de fracture numérique, même en haute zone aujourd'hui, on a la fibre sur tout le département. Même en haute zone. 539 communes, 230 000 habitants, il n'y a pas plus rural comme département, il y a la fibre partout. Donc, n'opposons pas les territoires ruraux aux territoires urbains. Aujourd'hui, on n'empêche pas les entreprises de travailler. n'empêchent pas les clients d'être livrés. La seule chose qu'on empêche et laquelle on s'est engagé ici le 14 novembre, c'est que ces entreprises ne puissent plus appeler ceux qui ne le souhaitent pas. Je vois pas ce qu'il y a de contrariant sur le domaine. En plus, je trouve que c'est un petit peu fort de café. À moi, président délégation des entreprises, sociolibérale mais plutôt libérale que sociale, Et je l'assume, je le maintiens cher Fabien, mais je l'assume de vouloir empêcher les entreprises de travailler. rien dans ce texte n'empêche les entreprises de travailler, absolument rien. Et puis la troisième raison, pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi sommes-nous des élus ? Pourquoi sommes-nous des parlementaires ? Est-ce qu'on l'est pour défendre l'intérêt général ou est-ce qu'on l'est pour défendre quelques intérêts particuliers ? Le sénateur Duplomb disait ce matin en commission, ça concerne trois voire quatre entreprises. Moi je vous pose la question, chers collègues. Est-ce qu'on est là pour répondre à la préoccupation dont on entend parler tous les jours de l'ensemble de nos concitoyens, de toutes les Françaises et les Français, du plus modeste au plus élevé ? et de ne pas respecter notre engagement et la parole qu'on a donnée. C'est vraiment les raisons pour lesquelles je vous demande, chers collègues, mais de la manière la plus sincère, la plus solennelle qui soit, de retirer vos amendements, de faire honneur au Sénat à votre engagement, ou de voter contre dans le cas où ils sont maintenus. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, comme votre avis est négatif, au nom de la Commission sur les amendements, logiquement, il ne peut être que négatif sur les sous-amendements. Tout à fait. Et donc vous engagez aussi la Commission sur les sous-amendements. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Donc les amendements 22 et suivants proposent enfin de créer une exception aux règles d'encadrement du démarchage téléphonique, encadrement qui est souhaité par les uns et les autres. d'ouvrir une dérogation, d'ouvrir une exception est toujours une brèche à un moment donné. Pourquoi telle exception ? Pourquoi tel secteur d'activité ? Pourquoi telle nature d'entreprise ? Pourquoi telle nature Au Au demeurant, c'est vrai que les produits qui sont cités ici, que sont les produits alimentaires ou d'animaux de compagnie, ne sont pas forcément les produits qui aient été cités ou ciblés dans l'esprit de cette volonté de modifier toutes les règles. d'encadrement du démarchage téléphonique, ce n'étaient pas forcément les principaux irritants dans le cadre de ces démarches. Il faut aussi indiquer que ce type de services de produits alimentaires qui sont livrés à domicile avec un dispositif de démarchage téléphonique répondent à des enjeux de territoire, à des familles, à des citoyens, qui n'ont pas forcément toujours la possibilité de se déplacer. En tout cas c'est un véritable service qui fonctionne très bien sur les territoires et peut-être plus sur les territoires ruraux. Donc c'est un élément à prendre en compte. Il y a également le fait que Un certain nombre d'entreprises ont construit, alors peut-être quelques-unes effectivement cela a été dit, leur modèle, un modèle économique sur cette base. Il faut tenir compte aussi de cette modification que l'on donne à un moment donné, il faut laisser le temps aux entreprises de s'adapter. Voilà, ça c'est un élément important. Moi je suis à la fois ministre de la consommation, donc attachée à tout ce qui concerne le démarchage téléphonique qui protège les consommateurs. Je suis également ministre des entreprises et je pense qu'on qu'on peut laisser le temps aux entreprises de s'adapter. Alors, si je suis défavorable sur l'amendement en tant que tel puisqu'il établit une dérogation qui n'est pas limitée et donc ça, ça ne me paraît pas possible parce qu'il y a une volonté très forte de répondre aux enjeux de démarchage téléphonique comme cela a été exprimé suite aux travaux du sénateur Verzelen. En revanche, je pense que l'on peut prendre en compte des situations particulières. Je pense que la situation économique de nos entreprises le mérite. J'avais à l'Assemblée nationale donné un avis favorable, un sous-amendement qui limitait cette dérogation à une période de 18 mois parce que ça me paraissait être un délai assez suffisant, normal, pour permettre à une entreprise de s'adapter. Là, le sous-amendement porte un délai supérieur, un délai de 60 mois, un délai de 5 ans, ce qui est quand même un délai important, donc ça me paraît un petit peu trop important par rapport aux besoins qu'une entreprise a de s'adapter, donc je mettrai un avis de sagesse sous les sous-amendements, et donc si les sous-amendements sont adoptés, adoptés, un avis de sagesse sur l'amendement. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Madame la Ministre, j'ai l'impression d'avoir parlé en l'air. Mais si, vous me dites Madame la Ministre, il faut comprendre les entreprises, il faut les laisser travailler, notamment sur les territoires ruraux, on a peut-être des personnes qui ont besoin, mais rien dans la loi n'interdit. Rien dans la loi n'interdit aux entreprises de continuer d'appeler, de prendre les commandes, de livrer, et rien n'interdit les consommateurs d'être livrés par les produits qu'ils entendent, comme ils l'entendent. quand vous dites derrière les territoires ruraux, les entreprises, faut les comprendre, etc., ben oui, mais elles sont comprises dans la loi, puisque tout est fait pour qu'elles puissent continuer de travailler. Ça, c'est la première chose. Après 5 ans, Dans 5 ans, on aura plus ni le même président de la République, ni les mêmes députés, ni une élection présidentielle. il n'y aura plus beaucoup de nous qui seront... Tous seront repassés à l'élection aussi. Tous les députés seront repassés aux élections. Enfin, 5 ans, ça veut dire... Excusez-moi, 5 ans, ça veut dire qu'on maintenait les tellement longs. que ça va devenir perpétuel. De toute façon, on n'ira pas au bout des cinq ans sans que des problèmes resurgissent et qu'on en reparle. Gagnons du temps. On ne peut pas décemment et qu'on en reparle. Gagnons du temps. On ne peut pas décemment donner une dérogation sur cinq ans. Et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'ensemble des bancs ici. Quand on parle de dérogation pour certaines entreprises, 5 ans, là on était sur quoi ? 18 mois, et sur 18 mois déjà on disait, oulala, rendez compte, il faut que la loi aille vite. Là il s'agit de protéger les consommateurs, de protéger les Françaises et les Français, ça ne peut pas attendre 5 ans. Merci, M. Chaise, pour une explication de vote. On n'a pas voté spécifiquement sur cet amendement, puisqu'on a voté globalement sur l'ensemble des amendements. Et je pense qu'en faisant ainsi, c'est plutôt les avis du rapporteur que les avis de la Commission qui sont au banc ce soir. Mais je respecte, c'est comme ça, c'est une question de méthode, mais je tiens à le dire aussi. C'est plus l'avis du rapporteur que l'avis de la commission. J'ai cru comprendre dans le débat qu'on a eu ce matin que l'avis de la commission n'était pas tout à fait aligné avec l'avis du rapporteur. Remettre en cause certaines dispositions. On est dans une période, et ce n'est pas mes collègues d'en face qui vont me dire le contraire, où on peut remettre des choses en en cause comme l'eau et l'assainissement, comme d'autres sujets, parce qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, dans la discussion, dans les échanges, on n'a peut-être pas fait tout à fait tout ce qu'il fallait comme il le fallait. Quant à défendre les entreprises, moi ce n'est pas défendre les entreprises qui m'intéressent, c'est défendre effectivement les habitants de notre territoire rural qui aujourd'hui ont besoin de ces services et qui souhaitent les avoir. Alors, effectivement, vous exprimez le fait que, globalement, ils peuvent continuer à travailler sur leurs clients, sur leurs fichiers clients, mais pas faire de nouveaux prospects pour pouvoir se mettre en place et trouver des nouveaux clients. Moi, je fais une proposition, puisque je comprends que 60 mois, ça soit effectivement beaucoup, je suis prêt à modifier le sous-amendement pour le réduire à 36 mois. ce qui permet de faire un pas donc de chaque côté et de trouver une façon de compromis qui répondrait à la fois à cette volonté de faire appliquer cette loi sur le démarchage qu'on a voté et sur lequel j'ai été d'ailleurs défenseur en laissant une petite marge de manoeuvre pour faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver. après, M. Cannevet, bon, tout le monde, M. Verzelaine, bon, j'avais eu un petit espoir, je me suis dit, je vais glisser une clôture de discussion, c'est raté, donc tout le monde pourra parler. Mme Roumanie, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai peur que nous soyons en train de mettre le pied dans la porte. En mettant cette exception là, on va mettre le pied dans la porte. On n'est pas en train de dire que les produits surgelés sont interdits à la distribution en ruralité. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Les clients qui existent resteront des clients demain. On a la possibilité de consentir à un démarchage téléphonique. On a cette possibilité-là aujourd'hui. Donc on n'est pas en train d'interdire la distribution de produits surgelés en ruralité. Ne nous trompons pas. Nous devons effectivement, je pense, légiférer pour l'intérêt général et non pour l'exception. Nous avons une loi qui a été votée à l'unanimité dans notre assemblée et quelques mois plus tard, nous sommes en train de mettre un pied dans la porte. Je pense vraiment que rien n'empêche la distribution et c'est quelqu'un du rural qui vous parle. Donc on a la possibilité aujourd'hui de se faire livrer des surgelés en ruralité, on le fera encore demain. Et qu'est-ce qui nous fait dire quand on a un appel téléphonique, et nous en avons tous tous les jours, qu'est-ce qui va différencier le 06 des surgelés du 06 d'un autre démarchage téléphonique ? Qu'est-ce qui pose des problèmes aujourd'hui ? Vous savez moi je suis passée à côté d'un accident de ma fille parce que j'ai pas reconnu le numéro et j'ai cru que je me faisais démarcher téléphoniquement. J'ai pas reconnu le numéro, j'ai pas répondu au téléphone et j'ai appris quelques heures après que c'était un problème à l'école et que la maîtresse dans l'urgence avait pris son portable et n'avait pas téléphoné de l'école. Voilà. Et ça on y est confronté tous les jours. Et moi je suis désolée mais j'ai pas envie de me poser la question de savoir si c'est un démarchage de surgeler ou si ma fille a un problème à l'école. Et je pense que ça, on peut tous y être confronté tous les jours. Et c'est pas une histoire de surgeler en ruralité. Je vous remercie. Merci madame Le Héro pour l'explication de vote. Merci monsieur le Président. Alors monsieur le rapporteur, vous nous soulignez le respect du travail des sénateurs versés. le sénateur Verzelen et de Olivier Richard et le vôtre également que je respecte. Mais je souhaiterais qu'on regarde aussi le respect du travail des salariés et des entreprises. Et permettre aux entreprises de s'adapter par un délai d'application, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tout à fait accepter. C'est aussi le respect des services rendus aux personnes âgées et aux personnes vivant au milieu rural et n'ayant pas la possibilité de mobilité. Vous indiquez la fracture numérique n'existe pas. Si elle existe, cette fracture numérique, malheureusement, et aussi ce qui s'appelle l'électronisme et la difficulté d'accès aux nouvelles technologies, c'est aussi une réalité. Je voudrais aussi rappeler que les députés ont voté à une très large majorité, ont approuvé à l'Assemblée nationale cette exception alimentaire. Donc je pense que c'est aussi un élément que l'on pourrait prendre en compte. Et quant au respect de l'intérêt général, et non le fait de répondre à des intérêts particuliers de quelques-uns. L'intérêt général c'est aussi tenir compte des particularités et des situations particulières et en tenant compte de ces particularités je pense que nous pouvons trouver une solution médiane qui permette de répondre à l'objectif du démarchage abusif mais en même temps de préserver et nos entreprises les salariés mais aussi les personnes qui bénéficient de ce service. Merci. Merci. Monsieur le Président, Gontard, vous avez la parole pour expliquer son vote. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai un peu du mal à comprendre le débat. J'ai envie de soutenir le rapporteur. Depuis que je suis tout petit, je vois le camion de congélateur qui arrive dans la cour de chez moi pour livrer ses produits. C'est un peu le quotidien quand on vit dans un village rural. Mais en fait, je n'ai pas l'impression que tout ça va être mis en cause. J'ai l'impression que dans ce que j'entends, c'est la fin de ces livraisons. Non, ça sera exactement la même chose. On aura toujours le camion qui va venir livrer. Il aura toujours la possibilité d'appeler ses clients, puisque c'est la possibilité qu'il a d'appeler ses clients pour savoir ce qu'ils souhaitent et prendre la commande tout simplement comme avant. La seule chose qui change, c'est le démarchage. C'est-à-dire d'interdire le démarchage et d'interdire que, alors que ce soit des entreprises de produits congelés d'autres, d'aller vers en fait et de pousser à la consommation mais rien n'interdira à une personne d'appeler et de faire venir ce son camion de congélation comme avant et puis ensuite il y a pareil cela la personne appellera c'est l'ensemble de ses clients donc j'ai un peu vraiment du mal à comprendre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui moi je trouve que Ce qu'a dit le rapporteur, elle est vraiment dans le bon sens. Et puis surtout, c'est que si on ouvre une brèche, comme il disait, je pense qu'on parle des produits de congélation. Pourquoi on ne parlerait pas d'autres produits ? On a aussi des produits d'autres grandes consommations et on sait que c'est très facile ensuite à... à prendre des biais donc moi je pense qu'on doit être très clair je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on veut plus de démarchage téléphonique donc voilà point et si on commence à faire des ouvertures ça ne marchera pas et après le fait de dire il faut laisser six mois cinq mois enfin peu importe

et interrogatif sur le vote que j'allais faire en séance. Parce qu'effectivement, on a tous dans nos territoires, et il n'y en a pas que trois, Olivier, on a on a tous des histoires, nous dans les Vosges, plus que dans les Vosges, c'est tiré. Enfin, on ne va pas les citer les uns après les autres. Si, peut-être. Président, on en a pour un certain temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est une réalité territoriale. Il y a un point que je voudrais corriger quand même puisque la région Grand Est est une des premières à être complètement fibrée. Ce n'est pas parce qu'on est fibré que pour autant on a une partie de nos concitoyens, hélas, qui sont en rupture et qui n'auront pas capacité effectivement d'utiliser la fibre et les messages, les mails pour faire des commandes. Donc le problème de la téléphonie reste entier. Moi j'ai beaucoup écouté notre rapporteur, je vais le suivre, je lui fais confiance, parce que dans l'explication qu'il a donné tout à l'heure, effectivement j'ai bien compris qu'on ne va pas empêcher celles et ceux qui restent dans cette dimension territoriale de proximité et il ne faut pas la négliger. N'oublions pas qu'on a passé le texte Madame la Présidente Egalime hier, qu'on se plaint parfois de la concentration de la distribution. Là, c'est une forme de distribution partagée territoriale de dimensions souvent départementales régionales. Et je pense qu'effectivement, notre rapporteur nous explique qu'on pourra continuer de le faire et surtout qu'on pourra continuer de faire de la prospé. Parce que ça, c'est essentiel. Si on ne peut pas continuer de faire de la prospé, ça veut dire qu'on signe tout simplement l'arrêt de mort des entreprises. Donc je fais confiance à notre rapporteur et je voterai contre ces amendements. Merci, monsieur Verzelen, pour l'explication de vote. monsieur le Président, mes chers collègues, peut-être expliquer quand même pourquoi ce sujet arrive. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on n'a pas parlé de ça il y a quelques mois, pourquoi on en est là ? Moi, si vous voulez, j'ai rien contre les entreprises ou les groupements d'intérêt qui prennent contact avec des élus quand un sujet les regarde. Là, en vérité, il y a une société où c'est hyper cavalier et c'est ni plus ni moins que du rentre dedans ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que le sujet est là. Et ce n'est pas toutes les entreprises du métier, d'ailleurs, je cherche à le préciser. Enfin, je le précise. Ensuite, Revenons sur les choses très concrètes. On dit à toutes les entreprises, avant de démarcher quelqu'un, tu vas, vous allez, allez obtenir un consentement. Et là, on dirait à ces entreprises, non, par des mots qu'on entend comme ça qui sonnent magiques, mais moi c'est pareil, je suis un hyper rural, territoire, rural, personne isolée. Mais très concrètement, donc on parle en gros de la petite dame qui est chez elle et qui est toute seule. Alors quand bien même elle est la fibre, peut-être qu'effectivement elle ne sait pas servir de l'ordinateur, on peut tous comprendre. Peut-être qu'elle sait aller ouvrir son courrier ou sa boîte à lettres pour voir de la pub. Peut-être qu'elle sait trouver un numéro au téléphone pour rappeler en disant j'ai envie de tel produit. Peut-être qu'elle a de la famille autour d'elle qui peut le faire. Et si elle n'a rien de tout ça, si elle n'a pas la famille, si elle ne sait pas ouvrir la boîte à lettres, si elle ne sait pas servir d'ordinateur et si elle ne sait pas appeler, il faut d'urgence que personne ne puisse s'appeler. Mais vraiment, que personne ne puisse la démarcher. J'insiste sur le sujet. Et 2.1, l'opérationnalité, ça a été dit. Si on met le pied dans la porte, d'autres s'engouffront dedans. Et pardonnez-moi, alors l'argument est peut-être simple, mais le rapporteur, dans sa discussion générale, prenait la métaphore de la route. C'est quand même particulier de dire, on dit à toutes les entreprises, on va rouler sur telle route à 100 à l'heure, et c'est pour tout le monde, si tu as une voiture verte et tel modèle, toi tu pourras rouler à 150. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas clair, et ça n'est pas exactement à la hauteur où on a eu du débat de tout le monde avant. Merci beaucoup. Merci monsieur Cannevet pour l'explication de vote. Merci M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues. Alors, ce débat est un peu surréaliste quand même parce que moi je crois qu'il faut qu'on tienne compte des réalités économiques dans notre pays. On a des entreprises qui, depuis plus de 50 ans, assurent de la livraison à domicile dans des territoires ruraux qui, bien souvent, sont des territoires excentrés. Alors je veux bien qu'on dise, ils pourront faire du prospect. Non, non, puisqu'à partir des moments où ils ne peuvent desservir que leurs clients, ça veut dire que le fichier client va se réduire petit à petit et que ces entreprises n'ont aucune perspective de développement alors même qu'elles emploient des centaines de salariés. Mais si. Mais si bien entendu, puisqu'ils ne pourront pas contacter les clients elles sont condamnées. Alors moi je veux bien qu'on remette en cause tout cela mais... La nécessité, c'est quand même qu'on laisse ces entreprises s'adapter, pouvoir s'adapter. Tout à l'heure, avant la pause, nous avons eu tout un débat sur un autre sujet où il fallait donner du temps concernant les RGE pour s'adapter. Nous étions un certain nombre à vouloir aller assez vite et puis non, on nous explique qu'il faut donner du temps. Et ici, lorsqu'il s'agit d'entreprises, Parce que là, c'est l'égalité de l'État. Mais lorsqu'il s'agit des entreprises, il faudrait que, justement, elles soient obligées d'obtempérer immédiatement. Mais ça n'a pas de sens. Enfin, on ne tient pas compte des réalités économiques. Et je crois que nous avons fait suffisamment d'erreurs par le passé dans l'examen d'un certain nombre de textes. pour se dire qu'il faut que l'on réfléchisse avant de mener des actions. Alors je crois qu'ici on serait bien inspiré quand même de réfléchir sur l'impact économique que cela peut avoir. Et l'impact économique qui sera particulièrement négatif parce que cela a été dit tout à l'heure, il y a encore un certain nombre de zones territoriales, les plus rurales, les plus excentriques, qui ne sont pas desservies par la fibre optique et qui donc n'ont pas des moyens modernes de communication. où l'appel téléphonique reste. Et si jamais la fraude venait de ces opérateurs-là, on l'aurait su depuis longtemps. Ce n'est pas le cas. Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le Rapporteur, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de me féliciter de ce débat entre nous. Et permettez-moi également de vous confier que je ne suis pas arc-bouté sur mon amendement. mon amendement. En revanche, il me semble possible d'envisager son retrait si nous consentons à voter les sous-amendements. Je répète, je ne suis donc pas arc-bouté sur ma position originelle. J'écoute ce qui se dit dans le débat. Je considère que faire aussi de la politique, c'est de rendre faisable le souhaitable et c'est cet objectif-là que nous essayons de poursuivre. Il ne s'agit pas dans mon esprit de remettre en cause l'objectif qui est poursuivi par cette proposition de loi. Donc dès l'instant, que l'on peut aménager le délai suffisant pour que les entreprises s'adaptent, eh bien, il n'y a pas lieu de maintenir mon amendement dans l'État où il est. Et il me semble, puisque l'idée des trois années ou des 36 mois a été évoquée, on peut très facilement converger là-dessus, non pas pour que la loi ne se réalise pas, mais pour la rendre pleinement efficiente. Merci de votre attention. Yannick Jadot soutenait le sous-amendement de M. Duplon en nous parlant de sa maman, voilà. Donc depuis ce matin, j'ai l'impression d'être dans le brouillard. Et le marin que je suis, c'est que dans le brouillard, il reste une chose essentielle, la boussole. À l'identique, non pas la corne de brume, la boussole. Pour savoir où l'on va. Comme l'a rappelé d'ailleurs, si justement cet après-midi, notre collègue Bernard Fialer, s'agissant de l'état de droit. Alors, je le dis au rapporteur, voilà, ce soir, ma boussole, c'est l'argument du rapporteur. Parce qu'il nous rappelle, au fond, la sagesse, le droit, la raison. Et je nous invite à à respecter cette raison. Et donc, en l'occurrence, nous retirons l'amendement de madame notre présidente Carrère. Très Très bien, monsieur Réchart, pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes en train là de nous interroger sur l'ouverture du démarchage commercial à la fourniture de denrées alimentaires et fournitures de produits pour l'alimentation des animaux. Je voudrais juste vous rappeler, mes chers collègues, qu'il y a dix minutes, ici, nous avons décidé, vous avez décidé, moi j'ai voté contre, d'interdire complètement le démarchage téléphonique dans deux autres secteurs. la rénovation énergétique, ça existait déjà et vous avez même décidé d'interdire dans la rénovation des logements pour permettre plus facilement l'adaptation aux handicaps ou ou en matière d'accessibilité. Mon cher collègue Bonvalet, moi je suis Je ne suis pas breton, je ne suis pas marin, je suis alsacien, mais moi aussi j'ai besoin d'une corne de brune. J'aimerais savoir dans ce brouillard où nous allons. Que va-t-il rester, mes chers collègues, de cette volonté d'un vote à l'unanimité rappelé par notre rapporteur pour précisément être tout à fait clair et dire que désormais on ne pourra plus, dans ce pays, démarcher sans l'accord préalable. des consommateurs. Je souhaite vraiment beaucoup de bonheur à la justice, parce qu'il y aura naturellement des contentieux, plein de contentieux. Tout à l'heure on a interdit, moi je suis persuadé que ça va tomber, on a interdit démarchage dans la rénovation énergétique. C'est contraire aux directives européennes, donc il y aura des contentieux, d'ailleurs on en a déjà perdu. Je l'ai dit tout à l'heure, tribunal administratif court d'appel. Mais comment la justice va-t-elle réagir avec comme ça des secteurs où les positions du législateur ne sont absolument pas les mêmes ? Donc franchement, moi je pense qu'il faut raisonner. Il faut raison garder et s'opposer clairement à ces derniers amendements. Déjà, je regrette que mon amendement tout à l'heure n'ait pas été retenu. Je vous ai dit qu'à mon sens, on va vers le plus en vue de contenue. Ça ne s'arrêtera pas si vous votez ça. Très court, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur. J'ai parlé d'un cas personnel, ma famille, puisque mes parents étaient commerçants ambulants. Ils distribuaient à peu près la moitié du département de la Côte d'Or. Et on a parlé tout à l'heure de Prospect. Et le Prospect, c'était pas la corne de brune, mais c'était le klaxon. Et ça marchait très bien. Donc je suis à vrai... l'avis du rapporteur. Alors, la corne de brune, le klaxon... Merci Monsieur le Président. Juste quelques mots pour dire que je vais aligner mon sous-amende demain à celui de mon collègue Laelegue et celui de mon collègue Chaz à 36 mois. Est-ce que je peux clôturer la discussion ? Merci. Il y a eu 11 explications de vote, je pense que c'est bon. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et ensuite Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne vais pas faire très long. Je vais juste répondre à une ou deux choses. Cher Michel Cannevet, mon vice-président à la délégation aux entreprises, je m'inscris en faux. Les entreprises pourront toujours faire de la prospection. C'est clair, c'est inscrit dans la loi. La seule chose qu'on leur interdit, c'est qu'elles ne pourront plus appeler les consommateurs qui ne souhaitent pas l'être. Mais ils pourront toujours faire de la prospection. Encore heureux. On comprend tous qu'un fichier client finit par diminuer un moment ou un autre. Et surtout, j'avais donné cet exemple-là en commission ce matin. Vous avez acheté, on parle de produits surgelés, un sachet de persil surgelé il y a plus de dix ans. Vous faites partie du fichier client. L'entreprise a le droit de vous appeler, même si ça fait dix ans que vous ne l'avez pas appelé. Par contre, le client a le droit de vous dire, à partir de maintenant, je ne souhaite plus être appelé. Et là, vous n'avez plus le droit de l'appeler. Ça ne peut pas être plus clair. Et un dernier point. Deux derniers points sur le temps qu'il faut donner aux entreprises. Mais la loi ne s'applique pas demain matin. Je crois qu'au plus rapide, la loi va s'appliquer début 2026, au mieux. Donc elle va avoir le temps de s'adapter. Et pour bien les connaître, je fais totalement confiance aux entreprises pour s'adapter à ce genre de modifications de loi. Je ne suis pas inquiet pour elles. le dernier point que je voulais citer, que je voulais répondre à notre collègue à Hellec, à Bernard Buie ou à Non, il a aligné son sous-amendement. Un autre collègue chaises, je ne vais pas être brutal, mais je le dis avec beaucoup d'amitié et beaucoup de considération pour vous, mais la parole donnée aux Français et aux Français le 14 novembre pour moi ne se négocie pas. On n'est pas sur un marché, on n'est pas en négociation commerciale, zéro dérogation, c'est le vœu que j'exprime et je reste dessus. Merci. Très rapidement, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé ce matin en commission des affaires économiques. Vous n'y étiez pas, et par rapport à ce que vient de dire Patrick Chaise, ce matin nous n'avons pas pu examiner en commission des affaires économiques les sous-amendements. puisque la séance hier s'est terminée plus tôt que prévu et ils n'ont pas pu être diffusés. On avait une commission à 9 heures, ce qui nous a amené simplement à dire et à suivre l'avis du rapporteur sur l'ensemble de ces amendements. Il n'y a pas du tout eu un flottement au niveau de la commission des affaires économiques. On a voté, on a discuté, on a discuté, mais on a voté et on a suivi le rapporteur. En revanche, On a bien dit que nous ne pouvons pas examiner les sous-amendements qui n'avaient pas été diffusés et publiés par la séance. On en débattrait ce soir en séance. C'est ce qui s'est passé mais la conclusion c'est que nous avons décidé de suivre l'avis du rapporteur sur les amendements et l'avis était un avis défavorable. J'ai entendu, cher collègue. Monsieur Faise, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous souhaitez corriger votre sous-amendement en faisant passer la durée de 60 mois à 36 mois, 36 mois, s'il vous plaît ? Je vous le confirme, M. le Président. Merci, M. l'Aélec. Vous faites la même correction ? Et M. Bué aussi, donc les trois sous-amendements 160, 174 et 175 deviennent identiques. Est-ce que je peux avoir l'avis du gouvernement sur ces amendements tels qu'ils viennent d'être rectifiés, Mme la Ministre ? — Sagesse. — Sagesse. La position de la Commission ne change pas, j'ai bien compris, M. le rapporteur. Donc je vais les mettre au voie qui est pour ces trois...

monsieur. Donc je mets au voie ces trois sous-amendements avec un avis défavorable de la Commission et un avis de sagesse du gouvernement qui est pour Merci. Qui est contre ? Ces sous-amendements ne sont pas adoptés. Nous passons donc ensuite aux, il en reste cinq, amendements identiques avec un avis défavorable de la Commission, un avis de sagesse défavorable J'ai compris. Donc deux avis défavorables sur ces amendements, qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. Et nous sommes sortis de cette discussion dans le brouillard, mais avec un phare. Voilà. Nous passons au 62, M. Losac. Losac. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je crains de voir se poursuivre ce débat enflammé. Mais l'objet de mon amendement rejoint ce que disait tout à l'heure madame la ministre lorsqu'elle évoquait ces entreprises ayant un modèle économique particulier et qui sont d'ailleurs prêtes à s'adapter dans un délai raisonnable. Parce que, qu'on le veuille ou non, il existe tout de même des spécificités professionnelles des secteurs économiques qui sont plus concernés que d'autres par cet article. Car ils vivent sur un modèle de commercialisation exclusif et concernant une démarche téléphonique, avec un appel justifié, raisonnable, hors de tout comportement désagréable et abusif. C'est le cas des EPV, les entreprises du patrimoine vivant, sur lesquelles je souhaite attirer votre attention, qui représentent des savoir-faire artisanaux et industriels tout à fait rares et tout à fait d'exception. avec plus notamment de 1000 structures et qui emploie près de 60 000 personnes. En effet, un très grand nombre de PME qui sont labellisés EPV Pour elle, la vente en direct, par le biais du démarchage téléphonique, du fabricant vers le client final et sans aucun intermédiaire, constitue l'unique solution commerciale. Alors effectivement, il s'agit très souvent de produits de luxe, mais des produits qui demandent très souvent un délai de réflexion, si je peux dire avant, la décision d'achat définitif. Et pour ce type d'achat, on a beaucoup d'entreprises qui s'astreignent à appeler une fois par an uniquement des prospects ayant préalablement exprimé, soit par courrier, soit par internet, leur intérêt pour tel vente, tel achat éventuel, pour tel objet d'art. Et je dirais que pour beaucoup de ces entreprises-là, qui sont très souvent des PME, des TPE, c'est vraiment une question de survie, une question de mort éventuelle pour ce type de société. Merci. Quel est l'avis de la Commission de ce rapporteur ? ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, chers collègues Lausac. Je pense que le moment qu'on vient de passer, vous n'aurez pas trop de surprise sur l'avis défavorable. Pas d'exonération, pas de dérogation, pas plus pour l'une que pour l'autre, donc un avis défavorable. Merci Monsieur le Président. Vous ouvrez ici une exception encore plus importante, beaucoup plus large que celle que nous avons exprimée il y a quelque temps, que vous avez exprimée sur les règles d'encadrement du démerchage téléphonique. Donc ça, ça me paraît être une dérégulation trop importante et par ailleurs elle n'est aucunement limitée donc ça n'est pas possible, ça ne correspond pas du tout à l'esprit de la proposition de loi et à l'esprit, à l'objectif de ce nouvel encadrement du démarchage téléphonique, donc avis défavorables. Merci, je mets au voie cet amendement 62 avec deux avis défavorables, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Monsieur Michel, vous présentez le 39 s'il vous plaît. Oui Monsieur le Président, Madame la Ministre, avec cet embandement, nous souhaitons une fois de plus renforcer la protection des des consommateurs, notamment face au développement de la sous-traitance, qui peut diluer les responsabilités et rendre plus difficilement identifiables les responsables à cas d'imperfection ou de défaut défaut de conception des travaux. Cet amendement vise ainsi à prévoir, parmi les mentions obligatoires devant être délivrées préalablement à la conclusion du contrat, l'identité de l'assureur du sous-traitant afin de faciliter les recours juridiques en cas de malfaçon sur les travaux. Par ailleurs, il arrive régulièrement qu'il y ait un changement de sous-traitant sur les chantiers en cours. La proposition de loi ne prouve rien sur ce cas de figure. Ainsi, il est proposé d'inscrire une mise à jour obligatoire du contrat en cas de changement de sous-traitant et d'en informer les particuliers, ceci afin de renforcer la transparence auprès des consommateurs. Merci. La vie de la Commission, monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Chers collègues Jean-Jacques Michaud, je sousquitte à l'objectif de votre amendement qui est de protéger les consommateurs. Mais la mise en œuvre risque de poser des difficultés aux entrepreneurs de bonne foi. Nous avons déjà précisé en commission qu'un contrat conclu sans information du consommateur concernant l'identité des sous-traitants et sans information du consommateur concernant les conséquences de la sous-traitance en matière d'aide financière était frappé de nullité. C'est déjà très fort. Si nous insérons l'obligation de transmission de l'identité des assureurs, cela sera une charge supplémentaire pour les entreprises. Vous connaissez mon goût pour la complexité. Je m'en éloigne et je m'en tiens très éloigné. Donc je vous demanderai soit le retrait, soit j'émettrai un avis défavorable sur votre amendement, chers collègues. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à flexifier un certain nombre d'obligations qui pèsent sur les professionnels et cela va à l'encontre de la simplification. Au demeurant, il y a deux éléments qui protègent aujourd'hui les consommateurs. Le professionnel avec lequel le consommateur a signé un contrat demeure le seul responsable des dommages ou des malfaçons qui sont liés aux travaux, même s'il y a des sous-traitants. Et deux, je rappelle que les organismes de qualification vérifient déjà la détention des assurances obligatoires par le professionnel avant de lui accorder le label RGE. Donc avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Je mets au voie cet amendement 39 avec deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Madame la Ministre, vous présentez l'amendement du gouvernement le 138, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement du gouvernement qui vise à préciser un certain nombre de modalités relatives au label RGE à l'agrément MAR. Un, cet amendement précise les modalités de suspension du label RGE et de l'agrément MAR en précisant que le caractère renouvelable n'est applicable qu'une fois. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait eu deux suspensions ne peut plus se voir renouveler le label et l'agrément. Deux, il réduit de 5 ans à 3 ans au maximum la période de carence qui pourra être prononcée par l'administration contre une entreprise dont le label RGE est retiré, durant laquelle elle ne pourra plus accéder au label, parce que ça nous paraît suffisant, une période de 3 ans. Et 3, elle élargit le spectre des motifs pouvant entraîner la suspension de l'agrément MAR, mon accompagnateur RENEV par la DGCCRF, en l'étendant notamment au manquement en matière de sous-traitance puisque, comme je l'ai répété il y a quelques instants, le professionnel est responsable de l'ensemble des dommages qui sont causés aux consommateurs et également des dommages qui sont réalisés par le sous-traitant. Voilà l'objet de cet amendement. sur le rapporteur ? Favorable, monsieur le Président. Favorable. Je mets au voie cet amendement du gouvernement avec un avis favorable de la Commission qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Monsieur le Président Gontard, vous présentez le 121, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le Président. Il s'agit dans cet amendement d'établir un délai de carence. délai de carence minimum d'un an après la suspension du label au signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l'octroi d'aide financière pour les travaux afin de renforcer la lutte contre la fraude aux aides publiques. Il s'agit d'une disposition qui avait été travaillée dans le cadre de la commission d'enquête sur les politiques de la rénovation thermique et c'est vrai que sur notamment le label RGE si on veut justement le conforter on a besoin de à la fois de mieux l'encadrer, de mieux le contrôler, mais aussi de sanctionner de manière plus lourde. Et le fait d'avoir un délai de carence minimum d'un an paraît utile, parce qu'on sait que des entreprises qui perdent leur label vont le retrouver très rapidement. Et donc, du coup, ça porte tout simplement tout simplement un crédit à ce label RGE. Merci. Merci. L'avis de la Commission de ce rapporteur. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, chers collègues Guillaume Gontard. La Commission en a fait introduit la possibilité pour la DGCCRF d'interdire à une entreprise dont le label a été retiré de recandidater au label dans la continuité des conclusions de la Commission d'enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique dont vous étiez vous-même rapporteurs. et que présidait notre présidente Dominique Estrosi-Sassonne. Il me semble pertinent de prévoir un délai de carence d'une durée suffisante pour que cela soit dissuasif. Je rappelle que nous avons précisé que cette sanction peut aussi s'appliquer aux personnes physiques afin d'éviter la multiplication de création d'entreprises. C'est vrai qu'on a fixé un délai maximum, une durée maximum de 5 ans, mais pas de durée minimum. Et donc je souscris totalement à votre amendement de fixer ces délais d'un an et donc un avis favorable sur votre amendement. Merci. Merci. L'avis L'avis du gouvernement, madame la ministre, s'il vous plaît. Alors cet amendement vient instaurer un délai de 4 ans de 3 années au plus alors qu'une durée maximale de 3 années apparaît enfin l'amendement du gouvernement qui vient d'être adopté il y a le 138 instaure un délai de 4 ans de 3 ans au plus et là vous proposez une durée simplement de 1 1 année pour verrouiller l'accès au marché ça me paraît insuffisamment dissuasif il faut laisser du temps il faut que la sanction puisse porter donc je vous demande un retrait pour faire en sorte que la durée de trois ans qui vient d'être adoptée à l'amendement précédent puisse être retenue, demande de retrait. Merci. Je mets au voie cet amendement 121 avec un avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement, qui est pour ? qui est contre, il est adopté. Monsieur Verzelen, vous présentez l'amendement 94, s'il vous plaît. Monsieur le Président, il vise à préciser que l'interdiction du démarchage téléphonique, enfin son encadrement, entrerait en vigueur au 1er janvier 2026. Monsieur le rapporteur, votre avis ? Favorable, monsieur le Président. Favorable. Madame la Ministre, s'il vous plaît, votre avis ? Alors, effectivement, il s'agit de la date, sachant que cet amendement revient sur la date du 11 août 2026. Alors, pourquoi avons-nous une date au 11 août 2026 ? Cette date correspond à la fin de la de la concession actuellement en cours pour la gestion du dispositif BlockTel et la résiliation anticipée de ce dispositif avec la société qui est en charge va générer une indemnisation relativement importante au profit du concessionnaire qu'on est valu aujourd'hui à près de 2 millions d'euros pour les finances publiques. Donc je pense qu'une distinction de huit mois et demi exactement, qui porte une valeur de 2 millions d'euros, c'est quand même assez important et je parle de ça devant la ministre en charge des comptes publics. Donc ça me paraît suffisant et par ailleurs ça laissera compte tenu d'un point qui a été évoqué pour l'adaptation des entreprises par rapport aux démarches, le sujet qui a été évoqué sur les entreprises qui livrent des produits alimentaires. Cela permettra d'apporter une réponse et de laisser plus de temps à l'adaptation de ces entreprises. Donc je suis défavorable à votre amendement pour aussi une question de finances publiques, parce que deux millions d'euros, ça n'est pas rien pour sept mois et demi. Sur un charte, vous avez de la parole pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, pourraient rencontrer des difficultés certaines pour faire évoluer leur modèle d'activité avant la date qui était prévue initialement, à savoir le 11 août qui, comme l'a dit madame la ministre, correspond à la fin du dispositif blocktail. Par exemple, les acteurs de la maintenance obligatoire, telles que par exemple monsieur le rapporteur, maintenance chaudière, maintenance voiture, climatisation et autres, démarchent souvent à intervalle régulier. et ne pourront recueillir le consentement de tous leurs contacts avant la prochaine échéance. L'anticipation de cette entrée en vigueur, pour moi, risque d'avoir des conséquences dommageables pour la vie économique, d'autant que, Madame la Ministre, je m'inquiète aussi sur l'apparution des décrets d'application qui pourraient, le cas échéant, ne pas être publiés dans les délais. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, par souci de sécurité et l'essai du temps, tout particulièrement au PME, moi je préférerais en rester à la date prévue, à savoir le 11 août. Oui, Monsieur le Président. Déjà deux éléments, le premier qu'on a un peu abordé. On a choisi de passer par un véhicule le plus rapide possible, c'est-à-dire le texte dont on parle aujourd'hui. Nous sommes en avril, si on vote ce soir, ça laisse quand même quelques mois. Il y a de l'attente chez les gens, je veux dire d'avril à août l'année prochaine. Tout ça me paraît quand même très éloigné. Je parle sur un plan politique et sur un plan de la perception. Ensuite, sur l'argument des pénalités block-tail. C'est un argument que j'ai du mal à entendre. Je vois pas pourquoi vous voudriez sortir de block-tail avant l'issue du contrat et payer les pénalités. Si j'étais taquin, je dirais que l'Etat paye block-tail depuis des années pour un service limité voire quasi nul. Donc laissez courir le contrat, qu'il aille au bout et vous embêtez pas avec les pénalités. avec les pénalités. Monsieur rapporteur, vous êtes à parole. Merci, monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, il faut qu'on soit un peu logique par rapport à ce qu'on a voté tout à l'heure. de la suppression, enfin de la limitation à deux rangs de sous-traitants à partir du 1er janvier 2026. Pour ça, il faut que la proposition de loi s'applique. Donc l'ensemble de la PPL doit s'appliquer au plus tard au 1er janvier 2026, y compris des articles concernant le démarchage téléphonique. Donc je maintiens et je confirme et j'insiste sur un avis favorable et je vous demande de voter l'amendement de notre collègue Huérzelen. Merci. Merci. Je mets au voie cet amendement 94 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre, il est adopté. Je vais mettre en voie la totalité de l'article 3 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous passons après l'article 3 à un un amendement et un sous-amendement. Monsieur le Président Gontard, vous présentez l'amendement 120, s'il vous plaît. Oui, merci monsieur le Président. Il s'agit aussi d'un amendement issu du travail de la commission d'enquête que nous avions réalisé effectivement avec la présidente Estrosi Sassone et qui souhaite obliger les sites internites et les publicités proposant des travaux de rénovation à inviter les particuliers à se reprocher d'une agence France Rénov'et également à inclure un lien de redirection vers la plateforme France Rénov'. C'est vrai qu'on s'aperçoit Aujourd'hui, si vous tapez « rénovation thermique » sur Internet, vous allez voir multiples multiples sites, plutôt souvent pour changer de chaudière, alors qu'on souhaite plutôt que les personnes aillent dans un vrai parcours de rénovation, soient accompagnées. le fait d'obliger l'ensemble de ces sites à pouvoir indiquer et mettre un lien sur ce site internet vers France Rénov'ça nous paraît tout simple et ça permet justement d'orienter dans la bonne direction les personnes qui se lancent dans un parcours de rénovation. Merci madame la ministre vous présentez le sous amendement du gouvernement 148 s'il vous plaît Merci Monsieur le Président. Ce sous-amendement vise à compléter un numéro de section et d'articles qui ne sont pas précisés dans l'amendement, renforcer les sanctions qui peuvent être prises et permettre leur modulation afin de dissuader les fraudeurs, créer une habilitation des agences et CRF pour relever ce manquement et renvoyer à un arrêté la définition des modalités d'information et leur contenu. C'est un sous-amendement pour rendre l'amendement pleinement opérationnel. Merci Monsieur le rapporteur. Votre avis s'il vous plaît. parce que fixer 7 500 euros, quand on voit certaines amendes que j'avais prévu de mettre, notamment sur le défaut des matriculations en registre national des entreprises, c'est autant. Je Je m'exprimerai par contre sur le sous-amendement de façon personnelle parce qu'il a été déposé après la réunion de la Commission. Donc sur le sous-amendement du gouvernement, Madame la Ministre, ça sera un avis favorable qui transformera mon avis sur l'amendement de notre collègue Gontard favorable sous condition d'adoption du sous-amendement, sinon défavorable. Merci. C'est très clair. Je vous remercie. Je veux mettre au voie le sous-amendement du gouvernement avec deux avis favorables qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Je veux mettre au voie l'amendement 120 tel qu'il vient d'être sous-amendé avec deux avis favorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Nous passons ensuite après l'article 3 à l'amendement 97, monsieur Monsieur le Président, il s'agit ici d'autoriser le filtrage automatisé des textos par les opérateurs et prévoir l'alignement du régime spécial au numéro de fixe sur celui qui est déjà applicable au numéro de mobile. Bien évidemment favorable Bien évidemment favorable Monsieur le Président. Favorable, je vous remercie Madame la Ministre, favorable également. Je mets au voie l'amendement 97 avec deux avis favorables qui est pour, qui est contre, il est adopté. Après l'article 3 Monsieur Verzelaine, vous nous présentez le 123 s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, et je vais en même temps parler pour les sous-amendements qui viennent, en tout cas que j'ai présenté, qui viennent derrière. Il y a quelques années, tout le sujet de la numérotation, de la classement des uns et des autres en démarchage ou en commercial a été confié à l'ARCEP. On a observé dans le temps des effets de bord, c'est-à-dire des entreprises ou des métiers qui ont été classés par la Recep avec la même numérotation qui est donnée pour des entreprises qui font du démarchage commercial. C'est un sujet que nous avions eu au Sénat ici, qui est revenu à l'Assemblée. Un, il y a le métier des sondeurs. et notamment des sondages à viser d'intérêts publics. Il est intéressant pour l'INSEE ou pour d'autres structures de savoir ce que les franchers mangent, comment ils se soignent, etc. Enfin, je crois qu'on voit de quoi on parle. Il y a le sujet de médiamétrie, notamment pour la radio et les mesures d'audience, qui aujourd'hui ne reposent sur aucun support technique, mais uniquement sur les appels téléphoniques. Et évidemment, s'il n'y a pas d'audience pour les radios, il n'y a pas forcément de la pub, et on perd de la pluralité de l'information. Un autre sujet est arrivé depuis quelques semaines, c'est celui du recouvrement des entreprises à qui il est confié d'aller chercher des factures impayées, qui eux aussi sont classées au même titre que ceux qui font du démarrage commercial. Or évidemment, c'est des gens qui sont déjà clients d'une société. Même la notion de consentement n'existe pas, mais c'est des effets de bord qui... qui les handicapent aujourd'hui dans leur activité. Donc ce qui apparaît aujourd'hui comme des sous-amendements, c'était l'idée de créer des exceptions, mais on est dans la ligne de ce qu'a dit le rapporteur, le but du jet de ne pas créer d'exception, mais c'était bien de mettre en lumière ces sujets-là. Donc je m'arrêterai à cet amendement 123 qui donne au ministre la possibilité de gérer ces sujets par arrêté et de décider qui sortira de cette numérotation. Et en plus, ce sera plus efficace auprès des opérateurs. Parce que si on fait une exception qui rentre dedans et qui ne rentre pas dedans, là si on gère par arrêté, on sait exactement qui aura le droit de faire des appels massifs et ceux qui n'ont pas le droit et que les opérateurs pourront couper. Je vous remercie. Merci. Je peux considérer que vous avez défendu les quatre amendements. — Alors vous pouvez considérer que j'ai défendu le 123 et que je retire les deux sous-amendements derrière. — Ce sont des amendements, c'est pas des sous-amendements. — Ce sont des amendements, pardon. — pardon. — pardon. — D'accord. Donc vous retirez le 100 et le 104, c'est ça ? Bien. Mais le 99, vous le maintenez. je me suis pris les pieds dans le tapis, je m'en excuse, je parle pas plus. Je maintiens le 123 et je retire le 99, et le 100. C'est compris. C'est Madame Gruny, vous voulez présenter votre amendement, s'il vous plaît, le 104 ? Je vais le retirer au profit des amendements de M. Verzelen, qui vient de défendre. Très bien, c'est clair. Monsieur le rapporteur, votre avis sur l'amendement ? 123, seul restant. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Merci à notre collègue Pascal Gruny Merci qui est 123, qui est d'une importance capitale pour ces entreprises qui sont aujourd'hui considérées et classées par l'Arceb comme des entreprises de démarchage mais qui ne font pas de démarchage. En revanche Madame la Ministre, je vous alerte sur la nécessité que cet arrêté inclut bien les sondeurs ou encore les entreprises de recouvrement de créances qui devraient avoir la possibilité de recourir à des automates d'appels sans pour autant être forcés d'utiliser des numéros que nous associons aujourd'hui à de la fraude. Et je souhaite que les décisions soient prises rapidement pour que l'ARCEP accède enfin à ces demandes de ces entreprises si importantes. Merci. Alors cet amendement présente un intérêt parce qu'il permettra finalement à un nombre très limité de professionnels et c'est aussi l'objectif qui sera défini par arrêter de pouvoir avoir recours à des automates d'appels sans pour autant devoir utiliser les numéros polyvalents vérifiés. Je pense par là en premier lieu à tout ce qui est enquête statistique et sondeur, ça a été évoqué ou d'autres destinés à la recherche scientifique. Aujourd'hui ces appels sont confondus par les citoyens avec le démarchage commercial et cette liste permettra d'apporter une réponse. J'ai entendu monsieur le rapporteur votre demande d'avoir un arrêté rapide, j'y veillerai. Tous les Tous les moyens pour répondre. J'ai entendu également votre demande par rapport au sondeur aux entreprises de recouvrement de créances. Je pense qu'il faudra effectivement prendre en compte toutes les catégories qui le nécessitent sans pour autant avoir une liste d'une exhaustivité exhaustivité importante puisque ça mettrait à mal finalement l'esprit de la PPL. Donc avis favorables. Merci, je mets au voie cet amendement 123, avec deux avis forables, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Après l'article 3, l'amendement 98, monsieur Verzen, vous avez la parole. cet amendement, il autorise expressément le partage d'informations, évidemment dans le cas d'une efficacité de l'action, entre les autorités concernées, la DGCCRF, l'ARCEP et la CNIL. Merci, qui est l'avis du rapporteur. favorable, l'avis du gouvernement favorable aussi. Je mets au voie l'amendement 98 avec deux avis favorables, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Monsieur le Président Gontard, vous présentez le 122, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, cet amendement pour des questions de recevabilité, on l'a transformé en rapport et sur la création d'une base de données. qui soit géré par l'ANA, intégrant les demandes d'aide, les chantiers de travaux et les contrôles réalisés au titre de la prime de transition énergétique et des certificats d'économie d'énergie. C'est un amendement qui a été travaillé avec la Confédération de l'Artisanat et des petites entreprises du bâtiment, qui paraît important si on veut justement avoir un suivi et une vraie réflexion et un vrai retour sur justement tous les mécanismes de fraude qui peuvent se mettre en place. qui est une vision croisée sur les différents types de fraudes et notamment leur évolution. Et ça nous paraît important d'avoir justement une base de données qui puisse être gérée par par l'ANA. Donc on l'a mise sous forme de rapport, mais c'est uniquement pour des questions de recevabilité. Merci. Monsieur le Président. Il existe déjà des partages d'informations, notamment entre l'ANA et le pôle national des certificats d'économie d'énergie. Je pense qu'aller vers la création et l'administration d'une nouvelle plateforme et d'une nouvelle base de données, ce serait une charge importante et redondante avec des dispositifs existants. Avis défavorables. Merci. Je mets au voie cet amendement 122 avec deux avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Mes chers collègues, nous revenons au cours normal de la discussion des articles. Il est bientôt minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin d'achever l'examen de ce texte. Si on continue à ce rythme-là, je pense qu'avant une heure du matin, nous aurons fini le texte. Nous passons donc à l'article 4. Bonsoir Madame la Ministre, vous avez la parole. Bonsoir Monsieur le Président. Nous revoilà parti donc sur la suite de nos dispositions qui ont trait au cœur de ce texte auquel nous avons maintenant la chance d'y avoir vu ajouter les mesures contre le démarchage. Cet amendement vise à fixer les seuils de franchise. du dispositif des C2E pour éviter des effets de contournement qui sont aujourd'hui constatés, notamment de la part des metteurs à la consommation de fioul et de carburant. Pour parler français courant, il s'agit ici de donner des précisions sur les conditions dans lesquelles sont fixés les seuils de franchise pour justement, je vous le dis, le fioul domestique et les carburants automobiles qui sont deux secteurs sur lesquels nous voyons qu'il nous faut être plus carrés. Merci madame la ministre, monsieur le rapporteur, l'avis du gouvernement ? Favorable monsieur le président. Je mets au voie cet amendement 137 du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Madame la ministre, vous continuez avec le 141 s'il vous plaît. Alors il s'agit de garantir la possibilité de contrôler, de sanctionner les opérations frauduleuses d'économie d'énergie en conservant les responsabilités respectives des acteurs du dispositif. L'enjeu c'est que nous puissions prévoir des niveaux de responsabilité du mandataire qui soient fixes, puisque au fond ce sont souvent des chaînes avec des apporteurs d'affaires dans une part et la fourniture de dossier clé en main parfois. il nous faut bien sécuriser qui est responsable de quoi, et que la dilution de la chaîne n'aboutisse pas à une dilution des responsabilités. Merci, qu'ait l'avis la Commission, ce rapporteur ? Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mes chers collègues, Madame la Ministre, votre amendement n°141 visa supprimer la définition des conditions de mandat par dépré en Conseil d'État. Une fois n'est pas coutume, je n'y serai pas favorable, pour deux raisons notamment. En premier lieu, cela reviendrait sur les travaux de notre Commission, puisque cette disposition a été introduite par un de mes amendements. Et en second lieu, les difficultés juridiques avancées ne sont pas avérées. Ça sera donc, je le confirme, un avis défavorable de la Commission. Merci. Merci. Je mets au voie cet amendement 141 du gouvernement avec un avis défavorable de la Commission, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement 144 n'est pas défendu dans l'hémicycle. Et ensuite, il y a quatre amendements identiques. Le 33 n'est pas défendu. Et nous passons au 48, M. Biac. Il est défendu. Je vous remercie. Monsieur Cannevet, pour le 56, défendu. Le 81, madame Nadie, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Si cette mesure est pertinente pour lutter contre la fraude dans les demandes des particuliers, elle risque de ralentir des projets industriels majeurs dont l'instruction est déjà complexe et longue. Allourdi en ces procédures irait à l'encontre des efforts de réindustrialisation et de simplification administrative. Nous proposons donc de préserver le développement de projets stratégiques tout en maintenant des contrôles adaptés. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces trois amendements identiques, Monsieur le rapporteur ? Merci Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Concernant ces trois amendements qui ont le même objet, ils visent à limiter la faculté de suspension de la procédure d'instruction des C2E aux seules opérations standardisées. Il ne me paraît pas opportun pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il ne tiendrait pas compte des travaux de notre Commission. En effet, l'un de mes amendements a permis de rendre la suspension de la procédure d'instruction facultative. Plutôt que de figer une automaticité rigide dans la loi, nous avons préféré renvoyer une appréciation au cas par cas dans le cadre de la mise en demeure du ministre chargé de l'énergie. C'est plus souple. Plus encore, il présenterait de notables insuffisances juridiques. D'une part, il érigerait dans la loi une distinction entre les opérations standardisées et les opérations spécifiques qui n'existent actuellement que réglementairement à l'article LR 221-13 du Code de l'énergie. il ne traiterait pas équitablement les particuliers, les collectivités ou les entreprises bénéficiant des C2E, selon qu'ils mettent en œuvre des opérations standardisées ou des opérations spécifiques. Cela complexifierait l'action administrative et générerait un risque contentieux. Devant toutes ces raisons, je vous signifie donc une demande de retrait, sinon ce sera un avis défavorable. Merci Monsieur le Président. C'est un avis de sagesse parce que je comprends bien l'idée de faire au fond porter uniquement la suspension sur les opérations standardisées et au fond de protéger les progrès des très grands industriels. Je vois bien la logique et j'en comprends la dynamique. Néanmoins comme le dit le rapporteur, je rappelle qu'on est là pour lutter contre la fraude et il n'y a pas que des opérations standardisées où il y a de la fraude. Donc il ne faut pas que la loi nous empêche, dans des cas où ce serait vraiment nécessaire de pouvoir suspendre, de le faire. Donc j'aime bien l'idée de se dire que c'est surtout pour les impérations standardisées de grande ampleur qu'on va suspendre, mais je préférerais qu'on garde l'option de pouvoir le faire dans des cas et des affaires plus complexes. Donc sagesse. Merci. Je mets au voire ces trois amendements identiques, 48 56 81, avec un avis défavorable de la Commission, un avis de sagesse du gouvernement qui est pour ? qui est contre, ils ne sont pas adoptés. Je vais mettre au voie la totalité de l'article 4, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article 4 est adopté. Nous passons ensuite à l'article 5, avec deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier est le 112. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Monsieur le Président. Cet amendement de notre collègue Jean-Baptiste Blanc propose de rétablir l'expérimentation du contrôle vidéo à distance supprimé lors de son examen en commission. Merci Monsieur Klinger. Monsieur Michaud, vous présentez le 44 s'il vous plaît. Il est défendu. Quel est l'avis du rapporteur sur ces deux amendements en discussion commune ? Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai une petite incompréhension sur votre amendement parce qu'il vise à rétablir l'expérimentation des contrôles visuels à distance, les CVAD, sur les C2E. Alors que cette expérimentation a aujourd'hui, ce dispositif a été aujourd'hui rendu pérenne. C'est rentré dans la loi. Donc pourquoi expérimenter quelque chose qu'on a rendu pérenne ? Voilà, donc demande de retrait ou avis défavorable. Merci. Merci, Monsieur le Président. La même chose. L'article 5 vient de dire qu'on allait le faire dans la loi, donc retrait, puisque je pense que votre démarche est satisfaite. Et on a même le luxe de ne pas devoir passer par une expérimentation. Oui, contrôler visuellement à distance la réalité. Voilà, donc merci beaucoup. qui vote contre, qui s'abstient. L'article 5 est adopté après l'article 5. Monsieur le Président Gontard, vous nous présentez l'amendement 118, s'il vous plaît. Oui, merci, monsieur le Président. Cet amendement, qui s'inspire également de la proposition numéro 9 du rapport de la Commission d'enquête sur la politique de rénovation énergétique, vise à conditionner les aides à la rénovation à un contrôle sur site durant le chantier. Il manque quelques instants quand même parce que ça me paraît être un amendement qui me semble important par rapport à tout ce qu'on a pu discuter jusqu'à présent sur la question à la fois des fraudes, sur la question de comment on peut faire écarter les entreprises peu scrupuleuses, sur les questions de travaux de rénovation. et on sait que notamment le label RGE n'est pas suffisant pour avoir une bonne qualité des travaux beaucoup de travaux qui sont réalisés qui en fait ne sont jamais réellement réceptionnés et qui laissent évidemment à désirer et notamment avec des entreprises peu scrupuleuses. Et là l'idée, et ça a été travaillé et c'est particulièrement demandé par la CAPEB et par les artisans du bâtiment de mettre en place un contrôle sur site à la fin du chantier et en fait c'est tout simplement s'inspirer de ce qui existe pour l'électricité avec le consuel qui est quelque chose qui fonctionne très bien où on a ce bilan en fin de chantier qui permet de qualifier la réalité des travaux mais aussi ça permettrait à des entreprises qui ne sont pas RGE et on sait qu'on a beaucoup d'entreprises de qualité qui ne sont pas RGE qui justement ne répondent pas à ce marché là et que c'est plutôt des entreprises de faible qualité souvent qui y répondent, de pouvoir justement se missionner sur ces chantiers et ça nous paraît important puisque en fait sans être RGE elles auront cette validation en fin de chantier et puis ça permettrait aussi justement si elle veut être qualifiée en RGE de dire qu'au bout de trois ou quatre chantiers sur lequel elles ont été, elles ont eu un avis favorable de pouvoir devenir entreprise RGE donc à la fois ça conforterait le label mais également ça permettrait à l'ensemble des entreprises de pouvoir missionner et surtout de les faire monter en compétence. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Quel est l'avis des familles La vie défavorable de la Commission, monsieur le rapporteur. le rapporteur. Quelle anticipation monsieur le Président ! C'est déjà indiqué, je l'ai. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cher Président Guillaume Gontard. Je ne serai pas favorable à votre amendement parce qu'il ne correspond pas réellement aux recommandations de la commission d'enquête sur la rénovation énergétique des bâtiments dont vous étiez vous-même le rapporteur et qui avait comme présidente notre présidente Dominique Estrosi-Sassonne. Cette commission d'enquête a proposé d'introduire un contrôle de type Conceal ou Caligase pour les travaux de rénovation effectués par des artisans pour qui le label reconnu Garand de l'environnement, RGE, n'est pas rentable ou trop complexe et ce pour simplifier et faciliter l'engagement de très petites entreprises. Sauf que là, dans votre amendement, vous voulez le généraliser à tous les travaux. Ce qui est vraiment tout autre chose. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai soit de retirer votre amendement, soit un avis défavorable, chers collègues. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, du gouvernement, Merci, Monsieur le Président. Même avis, parce que je comprends la logique de vouloir se dire, au fond, la meilleure lutte contre la fraude, c'est le contrôle systématique. Mais moi je ne sais pas et je ne crois pas que nous ayons les moyens de contrôler 53 000 entreprises et 100% des chantiers. On voit bien qu'il y a, et d'ailleurs ce serait lancer une suspicion sur l'ensemble de ceux qui travaillent bien. Je pense qu'on a plutôt besoin d'avoir des outils de repérage, des outils par la repérage fiscale, par le repérage des pratiques bancaires, par le repérage d'éléments que nous repérons. Tous effectivement, avec maintenant une plus grande faculté, contrôler 100% des chantiers. Je vous le dis, nous n'en avons ni les moyens ni les effectifs. À court terme, il me semble que ce serait en fait le mettre dans la loi, je crois nous créerait une très grande fragilité de capacité de mise en oeuvre donc je ne suis pas favorable à votre amendement monsieur le sénateur merci monsieur le président gontard pour l'explication vote Là, on ne s'adresse pas à l'ensemble des travaux, on s'assemble aux travaux qui, justement, auront des subventions dans le cadre de la rénovation énergétique et la rénovation thermique. Pour répondre à madame la ministre, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord, un, ce n'est pas de la suspicion sur les entreprises puisque c'est demandé par les entreprises. C'est une demande très forte et depuis très longtemps par la CAPEP, par les entreprises du bâtiment et par les petites entreprises du bâtiment. bâtiment. pour garantir parce qu'en fait elles n'ont aucun souci puisqu'elles sont en général et à 90-95% de très bonnes entreprises en capacité de faire les travaux et donc elle c'est pas un problème pour qu'il y ait une vérification en fin de chantier. Ensuite vous me dites c'est pas possible à appliquer. Ensuite, il suffit d'aller un petit peu sur un chantier. Vous avez divers dispositifs. Je redonne l'exemple du consuel pour l'électricité, quelque chose d'assez simple, qui n'est pas d'ailleurs une vérification systématique, le consuel. Une entreprise d'électricité ne va pas être contrôlée à chaque fois, mais on sait que quand elle est dans un cycle et quand elle a déjà répondu à certains nombres de choses, il y a quand même un bureau de contrôle qui atteste que les travaux ont été correctement réalisés. Moi je pense que c'est oui quelque chose qui se met en place, qui peut s'organiser, mais qui me paraît essentiel, qui me paraît essentiel justement si on ne veut pas que de l'argent public soit gaspillé, parce qu'on sait aussi très bien que dans la rénovation thermique, que ce soit de changement de chaudière sur du simple geste, sur des menuiseries, qu'on a des vrais problèmes de réalisation, de bonne mise en oeuvre. Et donc ça profiterait non seulement aux entreprises, ce que je disais aussi pour faire monter en gamme les entreprises, mais aussi ça les sécurise, et ça sécurise aussi certainement les entreprises qui font du travail de qualité, et notamment plutôt les artisans et les petites entreprises du bâtiment. Merci. Merci monsieur Blanc pour l'explication de vote. dans la continuité de ce que vient de dire Guillaume Gontard, on l'a évoqué, le sujet c'est l'efficience des aides, c'est la capacité des aides publiques à faire effet levier et de lutter contre les effets d'eubène qui ouvrent la porte effectivement à la fraude. On a évoqué à plusieurs reprises le fait qu'un certain nombre d'aides ne touchent pas leur cible. On a évoqué à plusieurs reprises, y compris pendant le PLF, le fait qu'il y ait des aides fiscales qui sont des aides au dispositif et non pas à la réalisation d'un ouvrage qui atteint une bonne qualité énergétique au niveau bâtimentaire. C'est ça le sujet et c'est à ça qu'il faut qu'on soit capable les uns les autres de mettre fin. C'est pour ça qu'on a eu un débat assez long sur l'article 3 terres C'est pour ça que dans ce cadre-là, à plusieurs reprises, on vous a demandé sur l'avis, sur l'amendement du gouvernement, quel était votre avis sur les dispositifs de contrôle à posteriori. Vous n'avez pas répondu. On repose ces amendements-là parce que, à mon avis, et c'est ce que vient d'expliquer le président Gontard, c'est voter cet amendement 118, c'est ce qui permet de faire sens et de donner de la pertinence à votre amendement sur l'article 3 terre, l'amendement du gouvernement, et donc faire en sorte que cette loi soit une vraie loi. S'il n'y a pas ça, encore une fois, un certain nombre de dispositifs qui ont été votés ne font que la loi par rapport à son objectif initial tombe. Madame la ministre nous a demandé la parole. Oui, merci beaucoup Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous avez raison sur un point. Nous avons des dispositifs qui parfois sont des objectifs de moyens et pas avec des outils où d'abord le résultat compte dans la modulation de nos aides. J'adorerais vous dire en tant que ministre des Comptes publics et surtout grande partisane de l'évaluation des politiques publiques que nous arrivons à mieux cibler nos dispositifs pour être sûrs que nous finançons bien des résultats et pas seulement des efforts. Ça c'est un point. Je pense que ce soir, minuit 16, sur ce texte, nous n'avons pas la matière et les éléments pour y arriver juste entre nous. Il y a néanmoins sur votre amendement, un point que je n'ai pas dit tout à l'heure mais qui est pour moi essentiel et qui génère et explique mon avis défavorable, c'est que vous proposez que l'entreprise contrôlée explique par quel organisme elle veut être contrôlée. Cette logique-là, comme la certification, comme le contrôle, c'est le... Oui, vous me dites, il y a des exemples qui marchent bien. Je peux vous dire que dans les cas dont on traite, c'est le cœur et le début de la fraude. Quand vous commencez à avoir des organismes de certification dont le capital est détenu par les organismes qui sont contrôlés et qui sont les certifiés, qui cherchent à être vérifiés, vous avez des montages extrêmement bien faits mais qui sont extrêmement fraudogènes et frauduleux. Donc voilà pour toutes ces raisons. Je pense qu'on peut probablement avancer parce que les questions structurelles que vous posez me semblent tout à fait pertinentes. Je ne crois pas que ce soit l'objet du texte de ce soir. Merci Madame la Ministre. Je mets au voie cet amendement 118 avec deux avis défavorables. Qui est pour Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Après l'article 5, Monsieur le Président Gontard, vous présentez le 119 s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le Président. Rapidement, puisque c'est, on va dire, un amendement de repli en fait, puisque par rapport à ce que vient de dire Madame la Ministre en disant qu'on ne savait pas comment faire, qu'on n'avait pas forcément de moyens en tout cas pour pouvoir le mettre en œuvre. Bon, je vous ai donné un certain nombre d'exemples et qui contredisent d'ailleurs réellement ce que vous venez de dire. Je rappelle par exemple sur les questions d'assainissement. C'est la même manière, on a un résultat sur site et c'est comme ça que les subventions sont versées, heureusement, et ça fonctionne très correctement. Voilà, c'est la même chose sur le constituel pour l'électricité, je pourrais vous donner d'autres exemples. Mais on a un dispositif qui existe, que vous avez mis en place dans le cadre de France Renov, qui est le DPE. Et ce DPE qui est un outil plutôt intéressant, sauf que le DPE n'est pas obligatoire à chaque fois que l'on va faire des travaux de rénovation thermique. Si on va changer sa chaudière, on n'a pas l'obligation d'avoir un DPE. Il me semble que pour moi, c'est nécessaire avant toute démarche, en tout cas de travaux de rénovation thermique, mais également d'avoir un DPE en fin de chantier, puisque ça permettra à la fois d'avoir, alors même si le DPE ne permet pas de voir la bonne facture des travaux, mais au moins vérifier en tout cas que ces travaux ont été réellement faits, et puis surtout d'avoir l'évolution de ce DPE et de cette catégorie de cette évolution dans la catégorie du bâtiment, ce qui permet quand même de vérifier que l'argent public que l'on met ne sert pas à rien. Et donc cet amendement propose un DPE avant et après chantier. Merci. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Président Guillaume Gontard. Encore une fois, mais vous l'avez dit dans cet amendement, vous reprenez des dispositions du rapport que vous avez réalisé au fin de la mission que vous avez réalisée avec la Présidente Estrosi Sassonne, mais vous l'avez modifié. Parce que dans le rapport vous parliez d'un DPE d'entrée, de manière à orienter, et on peut en convenir, au mieux les Français sur le bon parcours de rénovation qu'ils pourraient réaliser au niveau de leurs travaux. Par contre, vous ne parliez pas d'un deuxième DPE en fin de travaux. Et la raison principale, notamment pour laquelle je mettrais une demande de retrait en avis défavorable, c'est qu'un DPE, le coût d'un audit énergétique, donc d'un DPE, s'élève entre 1000 et 1500 euros, fois 2, on est entre 2 et 3000 euros, je trouve que la somme est quand même abusée. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Merci. Merci. Quelle Quelle est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre ? Merci Monsieur le Président. Si je faisais de l'humour, que certains pourraient considérer comme déplacé. Deux diagnostics, c'est deux potentielles sources de fraude. Pourquoi je dis ça ? Nous avons, avec Valérie Létard, mené dans les dernières semaines et derniers mois, un exercice très musclé, de reprise en main d'un certain nombre de diagnostiqueurs, qui vous le savez, organisaient fraude et corruption. Le particulier payait au départ pour avoir une très mauvaise note, pour ensuite faire des travaux qui allaient l'amener à une très bonne note, et payait à la fin pour que la note soit encore meilleure que la réalité. Donc je ne crois pas qu'on ait les moyens aujourd'hui de faire des DPE au départ et à la fin. On veut des bons DPE une fois, qu'on sache où on part. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, qu'il y a une location, il y a à nouveau un diagnostic. Donc en fait, les biens immobiliers, ils vont être constamment maintenant diagnostiqués. Mais je pense que l'enjeu, ce n'est pas de faire des diagnostics tout le temps, c'est de faire des bons diagnostics d'une part. Ensuite, effectivement, on pourrait avoir une logique. On fait avant, on fait après et on est financé sur la différence. Certains proposent ce genre de mécanismes. Nous ne sommes pas mûrs pour le faire et donc je suis défavorable.

moi j'y crois au DPE, je pense qu'il y a des évolutions à faire de dire qu'effectivement il est mal géré et que c'est source de fraude. Je pense l'inverse, je pense qu'on a l'encadré. Je rappelle qu'on avait déposé d'ailleurs un amendement pour une carte professionnelle. que vous ne souhaitez pas, je trouve qu'au contraire, on doit faire monter en gamme et professionnaliser sur les diagnostiqueurs. Ça c'est une réalité, mais alors allons-y et faisons-le. Et je pense qu'on ne peut pas dire à la fois, le DPE ne sert à rien, il n'a aucune utilité, et pourtant en faire le point central de nos politiques de rénovation thermique et énergétique. Donc voilà, et moi je pense que quand on réalise quelque chose, c'est bien de savoir d'où on part et où on arrive. Et moi, c'est ça l'utilisation claire et justifiée de l'argent public, de savoir à quel moment, de quelle qualité notre bâtiment est, vers quoi on va le faire aller. Et puis parce qu'on a besoin d'avoir une visibilité de notre parc immobilier. Si vous ne faites pas ça sur les copropriétés, je ne sais pas comment vous allez avancer. De ne pas avoir cette visibilité globale de l'avancée des travaux qu'on fait, pour moi, c'est mettre de l'argent public par les fenêtres. Si j'ai bien compris, puisqu'on arrive au terme de l'examen de cette PPL, on est en train de ressortir, si vous maintenez votre avis, avec la possibilité de conserver le fait que des plateformes de bricolage, par exemple, puissent faire depuis Paris des devis pour des travaux qui seront réalisés à 800 pour installer une pompe à chaleur, sans qu'on sache à un moment donné si ça a une efficacité ou pas sur l'amélioration énergétique du bâtiment. Je le dis, je pense qu'on loupe le coche. qu'on loupe le coche. Merci. parole. Merci, Monsieur le Président. Précisément non, Monsieur le Sénateur. Nous avons voté il y a quelques heures maintenant un article amendé d'ailleurs par le rapporteur, disant que pour ces acteurs qui ne sont pas eux-mêmes des professionnels du bâtiment, nous voulions créer un label qui soit une forme de qualité Et précisément dans ce label, non dans ce label nous allons dire quoi ? Qu'évidemment vous ne faites pas des devis à distance, les yeux fermés à 800 km. Et que quand vous êtes une plateforme de bricolage installée dans un département, vous ne pouvez pas proposer des devis pour des gens qui sont dans une autre région ou à l'autre bout de la France. Et vous savez quoi, les professionnels du bricolage ils y sont prêts, ils ne veulent pas imaginer ce genre de fraude et c'est bien pour ça qu'on vous a proposé les uns et les autres de nous donner un tout petit peu de temps jusqu'en 2027 c'était la proposition du rapporteur pour que nous ayons le temps 1 de définir la norme de qualité et de tester la manière dont, et bien je crois non pas seulement les marques mais potentiellement d'ailleurs les enseignes ou un certain nombre de professionnels locaux pourront assurer la tenue et le respect de ce label et de cette qualité sans être eux-mêmes des professionnels du bâtiment. Je pense que si vous avez des doutes, et bien nous mettrons aussi dans le label, je me tourne vers mes équipes, les éléments d'évaluation du dispositif, les indicateurs d'évaluation, Non, ça existe monsieur un certificateur de label, c'est précisément ce qui existe et qui aujourd'hui fonctionne plus ou moins bien. si on parle des grandes enseignes du bricolage, je pense que nous avons tout à fait les moyens d'organiser les choses intelligemment et de manière fiable. et de manière fiable. Merci Madame la Ministre. Je mets au voie cet amendement 119 avec deux avis défavorables qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Je vais mettre au voie la totalité de l'article 6 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, l'article 6 est adopté. Je mets au voie la totalité de l'article 7 qui est pour, Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'article 7 est adopté. À l'article 8, je suis saisi de deux amendements identiques. Le premier, celui de M. Michaud, c'est le 42. Vous avez la parole. Oui, M. le Président, Mme la Ministre, cet amendement a été proposé par Enedis, en effet les gestionnaires de réseaux publics d'électricité constantes. En effet, une forte augmentation du nombre de fraudes à l'électricité et la tendance va en s'aggravant. Or, les détériorations et les fraudes au compteur communiquants qui se multiplient sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l'ensemble des usagers des réseaux de distribution d'électricité via l'augmentation N18 du Turp. À ce jour, ces fraudes peuvent faire l'objet d'une sanction pénale. Toutefois, cette réponse pénale est souvent lente à se concrétiser en raison de la longueur des procédures devant le tribunal correctionnel et ce alors même que ces fraudes se multiplient. Cet amendement vise donc à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution le pouvoir de prononcer des contraventions

Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Concernant ces deux amendements de notre collègue Annick Jacquemet et du collègue Michaud, ils sont satisfaits. J'y ai veillé moi-même par un amendement que j'ai déposé en commission et qui a été voté et qui a modifié le texte. Donc étant satisfait, j'ai même été plus loin parce que j'ai intégré les compteurs gaz. Donc je suis allé plus loin. Donc satisfait et encore plus que satisfait. Donc je vous demanderai le retrait à défaut, en avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Alors, Alors, défavorable sur les deux amendements 42 et 2 rectifiés. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je peux d'ores et déjà annoncer un avis de sagesse sur l'amendement du rapporteur. L'intention d'éviter les fraudes aux compteurs, qu'ils soient électriques ou de gaz, est bonne. Il nous semble à ce stade un peu compliqué de donner des pouvoirs presque de polis judiciaires à des entreprises privées. Mais il y a l'idée qu'il puisse y avoir, au fond, résorption à l'amiable, voire amende, d'une certaine manière, pour les constats de fraude dans le cas de compteurs frauduleux. Donc sagesse, parce que je trouve que c'est une bonne idée, qu'il faut qu'on arrive d'ici, probablement la CMP, à voir comment rédiger pour que ce soit constitutionnel, ce qui n'est pas une mince affaire, mais on va le faire. Merci beaucoup. Merci, je mets au voie, oui, M. Canlevet, vous avez la parole. Merci, Merci, monsieur le Président, madame la Ministre, chers collègues. Alors, on va le retirer, l'amendement, mais je dis simplement que ce n'est pas la peine que la justice soit engorgée de procédures qui n'ont pas lieu d'être. Je le retire après avoir entendu les explications du rapporteur. c'est clair qu'aujourd'hui ce sont des agents qui sont assiamentés et qui donc découvrent des vols d'électricité en quelque sorte et il paraît légitime que cela puisse être sanctionné sans que des délais extrêmement longs et que la justice ait à voir ses affaires. Monsieur Michel, vous le maintenez ? Vous le maintenez. Donc je mets au voie cet amendement 42, avec un avis défavorable de la Commission, avec un avis de sagesse du gouvernement, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Nous passons ensuite à l'amendement 152 de la Commission, avec un avis de sagesse du gouvernement. Vous le défendez, monsieur le rapporteur ? Il est rédactionnel. Je mets au voie cet amendement 152, avec un avis de sagesse du gouvernement, qui est pour ? qui est contre, il a adopté. Je mets au voie la totalité de l'article 8, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article 8 est adopté. Après l'article 8, je suis saisi d'un amendement 131 du gouvernement. Vous avez la parole, madame la ministre. parole, madame la ministre. Nous en avons parlé tout à l'heure lors de la présentation d'un amendement de la sénatrice Goulet. Il s'agit de permettre l'accès au Répertoire national commun de la protection sociale pour les agents des services consulaires. Vous êtes un résident à l'étranger, vous souhaitez bénéficier d'une aide sociale ou d'une bourse scolaire. Pour cela il convient qu'aucune prestation ne vous soit versée en France et bien pour que l'agent consulaire puisse constater que c'est le cas il faut qu'il ait accès à la base de données qui regarde quelles sont les prestations sociales auxquelles vous avez droit ou pas. C'est pour passer du déclaratif au contrôlé et je pense que vous me suivrez mesdames et messieurs les sénateurs sur cet amendement. Merci monsieur le rapporteur, la ville de la commission s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Non seulement ce sera un avis favorable sur cet amendement, mais également sur les deux suivants du gouvernement Monsieur le Président. Très bien, je vous remercie. Je mets au voie cet amendement 131 du gouvernement avec un avis favorable de la Commission qui est pour, qui est contre, il est adopté. Nous passons au 140 du gouvernement avec un avis favorable de la Commission. Au but, il s'agit de permettre dans le cadre du compte personnel de formation que des suspensions de paiements formulés par d'autres administrations de contrôle s'imposent à la caisse des dépôts et consignations. Bref, s'imaginer qu'une administration découvre que telle entreprise est frauduleuse dans sa capacité à offrir des formations, et bien cet amendement permet que, automatiquement, la caisse des dépôts procède à la suspension des paiements. Là aussi, efficacité, dialogue entre administrations. Je crois qu'on est au cœur de ce que nous cherchons à faire depuis tout cet après-midi. Merci. Je le mets au vote. L'amendement 140 du gouvernement avec un avis favorable de la Commission, qui est contre. Il a adopté l'amendement 139 du gouvernement. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Il s'agit de renforcer l'efficacité des contrôles de l'IGAS, de l'IGF quand ils sont en cause des financements publics et de l'inspection générale de l'enseignement supérieur et de la recherche quand il s'agit d'établissements de formation. Je l'ai dit tout à l'heure sur un autre amendement, mais il est surtout présent ici. Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Ces inspections ne peuvent contrôler que les filiales ou bien les têtes de réseau, l'un ou l'autre. Plutôt les têtes de réseau. Et nous voudrions que les inspections puissent aller dans les filiales, c'est-à-dire dans les lieux où s'opèrent réellement les missions et n'est pas qu'un contrôle administratif ou fiscal ou comptable, mais bien des contrôles de terrain, et semble assez logique que nous le permettions, mais un petit article législatif le permettrait de manière automatique. Pardon, monsieur le Président, c'est ce qui s'est passé sur le contrôle des crèches. sur le contrôle des maisons de retraite. C'est ce que nous faisons actuellement sur les centres de formation. Mais nous avons beaucoup de mal à le faire à l'échelle des réseaux puisque les missions d'inspection sont a priori surtout fiscales et comptables et nous voulons aller voir ce qui se passe sur le terrain. est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Merci. Je mets au voie cet amendement 139 du gouvernement avec un avis favorable de la Commission qui, pour, qui est contre, il est adopté. Nous passons à l'intitulé et deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le premier, le 1, rectifier Quater, M. Canavette, vous avez la parole. il s'agit simplement de dénomer différemment le titre de la proposition de loi puisque Il s'agit d'inclure dans le titre diverses dispositions de lutte contre la fraude aux aides publiques car, à notre avis, le travail reste encore incomplet. Il y a encore beaucoup à faire. C'est dire que nous franchissons une étape par ce biais, mais loin de lutter véritablement contre la fraude aux aides publiques. Merci, M. Grosvalet. Vous présentez le 45 Rétif Equataire, s'il vous plaît. Oui, je vous ai invité dans la discussion générale à la sobriété. Donc il s'agit d'abord de ne pas tromper nos concitoyens, de dire ce qu'est cette loi, c'est-à-dire cette proposition de loi, un progrès, mais de ne pas dire ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga de la lutte contre les fraudes aux aides publiques. Quel est l'avis de la Commission, ce rapporteur ? Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Une proposition de loi ne pouvant avoir qu'un seul titre et qu'un seul intitulé, nous revient de choisir entre deux. Non mais sérieusement, Je demanderai le retrait de l'amendement n°1 de notre collègue Nathalie Goulet en faveur de l'amendement de notre collègue Grosvalet. Ça a été relevé notamment par Fabien Guay, ça a été relevé par vous cher collègue Grosvalet et par d'autres. On ne peut pas se contenter de dire toutes les fraudes. Dès l'instant on ne traite pas toutes les fraudes mais une partie des fraudes. Et donc je mettrai un avis, une demande de retrait ou un avis défavorable sur l'amendement numéro 1 et un avis de sagesse plutôt favorable à l'amendement de nos collègues Philippe Grosvalet. Merci. Je ne sais pas si j'ai le droit de ne pas donner d'avis, mais je pense que c'est une prérogative qui vous est pleinement souveraine. Il s'agit d'une proposition de loi. Ce n'est pas le texte du gouvernement. Il a été écrit par Thomas Cazenave. Il avait un titre qui reflétait le travail que Thomas Cazenave a mené. Nous en avons fait un peu plus ce soir. Donc si vous choisissez, je choisis de m'en remettre à vous, monsieur le rapporteur, pour l'excellent travail qui a été fait ensemble et pour vous remercier. Toutes et tous du soutien que vous donnez à nos administrations de lutter contre ce qui mine le pacte républicain, à savoir la fraude. Alors, Mme la ministre, votre choix va être facilité par le fait que l'amendement à rectifier Quater est retiré, donc il n'en reste plus qu'un. Voilà. Et j'ai compris que vous émettiez un avis de sagesse sur cet amendement. Donc je vais mettre au voie l'amendement 45, avec un avis favorable de la Commission de l'avis de sagesse du gouvernement, qui est pour le titre de la proposition de loi devient proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques. Je veux mettre au voix l'ensemble de cette proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote ? Monsieur Blanc, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. On a effectivement à travers l'examen de ce texte adopté un certain nombre d'avancées pour un meilleur ciblage, pour améliorer la lutte contre la fraude. Mais il y a aussi, et il faut le dire de manière très claire, un certain nombre de régressions qui apparaissent à la suite de cet examen. Je veux en citer quelques-unes. Premièrement, sur la question des étrangers, il y a une aversion de ce qu'il faudrait faire à nos yeux. Il y a aussi sur l'extension des pouvoirs de l'IGA, un certain nombre de mesures qui ont été adoptées sans étude d'impact et sans avis de la CNIL, cela nous interroge. Mais surtout, deuxième point, sur les aides. Là où on avait, et on vient d'en parler, un label simple, celui RGE. et la possibilité de s'appuyer sur celui-ci. Nous ressortons de ce texte avec la création d'un nouveau label, notamment pour les entreprises commerciales. Bonjour la simplification. Bonjour la simplification. Ce que nous demandent les entreprises du bâtiment, et nous avons travaillé avec celle-ci un certain nombre d'amendements, qu'il s'agisse de la FFB, de la CAPEB ou d'autres, c'est de la stabilité. C'est d'arrêter d'avoir des règles qui changent tous les six mois, à plusieurs reprises, notamment sur ma prime rénov', elles nous ont dit, mais attendez, A chaque fois qu'il y a un texte fiscal, les choses bougent. Si on veut

Il faut qu'on donne davantage de souplesse aux entreprises sérieuses, qu'on leur donne la possibilité de mieux travailler. Aucune des mesures que nous avons proposées pour nous assurer de l'efficience des aides publiques n'ont été retenues. Enfin, je veux le dire, nous ne partageons pas le calendrier de report à 2028. Je crois qu'il y a là un certain nombre de mesures, certes, qui vont dans le bon sens, un certain nombre de mesures techniques, notamment pour essayer de décloisonner. Tout cela est intéressant et important. Par contre, et pour conclure, l'objet, sur les trois points qui font l'objet de l'objet de ce texte, il y a des régressions que nous ne partageons pas. Merci, cher collègue. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote ? Je n'en vois pas, madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Je reprends très calmement la parole parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas vécu le même débat. Les étrangers, il n'y a rien dans ce texte qui est contre, ou pour, ou neutre. Il y a une communication entre les organismes de protection sociale et les préfectures pour que les organismes de protection sociale puissent demander si des pièces d'identité de vous, de moi, de nous tous, de vous de ne puissent être un vérifié comme valable et si elles sont frauduleuses qu'elles puissent être annulées. Je ne vois pas en quoi nous parlerions ici de quoi que ce soit sur le droit des étrangers. Nous parlons ici du droit des pièces identité. Deuxième élément, l'IGA, vous n'avez pas voté cet amendement ? Donc vous me dites qu'il n'y a pas d'études d'impact. Effectivement, il n'y en avait pas. D'ailleurs, pour cet argument, vous n'avez pas suivi le gouvernement. Vous êtes souverain. Ce n'est pas présent dans le vote que vous devez désormais réaliser. En 2028, vous avez choisi le sous-amendement du rapporteur qui porte à 2027. Donc je ne vois pas où est la régression. Et enfin, il n'y a pas de changement pour les artisans RGE qui sont honnêtes. Les seuls qui vont voir des changements, ce sont les frotteurs. Ce sont les fraudeurs, les artisans honnêtes par ce texte. Il n'y a rien qui change pour eux. Rien. Les seuls pour qui potentiellement cela pourrait changer, les seuls pour qui ça peut potentiellement changer, je pense en certifiant d'ailleurs leurs pratiques, ce sont les plateformes de bricolage qui pourront faire faire des devis dans un cadre organisé. Vous êtes aujourd'hui un artisan RGE en Haute-Saône, en Aisson dans mon département ou quoi que ce soit ailleurs dans le pays, dans la Somme ? Rien ne change pour vous. Vous êtes honnête, rien ne change. Donc je préfère qu'avant le vote, vous ayez, messieurs et mesdames, les sénateurs et sénatrices, une vision exacte de ce qui est mis au vote ce soir. Parce que sinon, quand j'entends régression, 2028, IGA étranger, on ne parle pas du débat que nous avons mené, je crois, avec beaucoup de sérieux et je crois beaucoup d'efficacité collective. depuis 16h30 aujourd'hui dont je suis je crois très fière. Au nom des équipes qui travaillent sur ces sujets, parfois je dois dire avec beaucoup de difficultés, du résultat obtenu. Merci madame la ministre, je mets au voie l'ensemble de la proposition de loi dont l'intitulé est ainsi rédigé. Proposition de loi renforçant la lutte contre les fraudes aux aides publiques qui est pour qui est contre, qui s'abstient à la proposition de loi et adoptée. Mes chers collègues, je vais lever la séance. La prochaine séance aura lieu le jeudi 3 avril à 10h30 pour l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifié en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale. La séance est levée.